J'informe le Sénat que des candidatures ont été publiées pour siéger au sein de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte commun sur la proposition de loi visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination.

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, chaque année, entre 40 000 et 50 000 personnes sont victimes d'une mort subite, souvent à la suite d'un infarctus, faute d'avoir bénéficié au bon moment de l'intervention d'une personne qui aurait pu leur sauver la vie en pratiquant les gestes de premiers secours et en relançant le coeur par un choc électrique, ou défibrillation, le temps que les secours médicaux interviennent. C'est pendant le temps que mettent les secours à arriver que l'état d'une victime s'aggrave ou que le décès intervient. C'est pendant ce laps de temps qu'il faut agir. Grâce à des gestes simples qui s'apprennent, chacun d'entre nous peut un jour sauver une vie ou éviter à une personne de lourdes séquelles. Ne rien faire, c'est de toute façon condamner la personne en arrêt cardiaque. Il est fondamental que toute personne témoin d'un arrêt cardiaque initie la « chaîne de survie » formée de quatre maillons qui procurent aux victimes d'urgences médicales les meilleures chances de survie : appel rapide aux services de secours et de soins d'urgence ; massage cardiaque entrepris rapidement défibrillation précoce en utilisant un défibrillateur automatisé externe ; soins médicalisés spécialisés rapides, rendus possibles grâce à l'appel au SAMU. La formation du public, et en particulier des jeunes, aux gestes élémentaires de premiers secours est une priorité pour le Gouvernement. La France, société de solidarité, confrontée à des menaces toujours plus présentes- catastrophes naturelles, accidents, attentats ... -, doit porter un programme ambitieux de formation aux gestes de premiers secours. Tout un chacun est confronté à des situations de détresse et savoir réagir permet de sauver des vies. Si des efforts très importants ont été mis en oeuvre pour initier ou former le public à tous les moments de la vie à la prise en charge d'une personne en arrêt cardiaque et à l'utilisation d'un défibrillateur automatisé externe, ou DAE, il reste encore du chemin à parcourir. Actuellement, on estime que seulement 20 % de la population française a suivi une formation aux gestes de premiers secours et que 50 % des élèves en classe de troisième ont bénéficié de la formation « prévention et secours civiques de niveau 1 », ou PSC1, alors que 80 % de nos voisins allemands et autrichiens sont formés. Les objectifs fixés par le Président de la République de formation de 80 % de la population aux gestes de secours sont inscrits dans le programme national de santé publique. Un travail interministériel piloté par le ministère de l'intérieur en concertation avec tous les acteurs est en cours afin d'en établir les modalités d'application. Une attention particulière sera apportée aux formations pour les jeunes générations, en fonction de leur âge : premier degré- dispositif « apprendre à porter secours » second degré- classe de sixième « gestes qui sauvent » et classe de troisième « PSC1 » ; enseignement supérieur- « rattrapage » des étudiants non formés au PSC1 et mise à jour des connaissances de ceux qui sont déjà formés. Dans ce cadre, l'arrêté du 30 juin 2017, cosigné par le ministre de l'intérieur et la ministre des solidarités et de la santé, a institué une sensibilisation aux « gestes qui sauvent » et défini le contenu et les modalités de la formation. Il convient maintenant de promouvoir cette formation. Cet arrêté prévoit notamment que les professionnels de santé peuvent dispenser la sensibilisation aux « gestes qui sauvent ». Le cadre réglementaire de l'apprentissage des gestes de premiers secours existe et se renforce. Le nombre de personnes formées augmente régulièrement, notamment chez les jeunes, mais il faut, mesdames, messieurs les sénateurs, dynamiser cette action en favorisant partout les initiatives visant à promouvoir l'appropriation de ces gestes dans la population. Depuis le décret du 4 mai 2007 relatif à l'utilisation des défibrillateurs automatisés externes par des personnes non médecins et modifiant le code de la santé publique, « toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe Il convient désormais d'encourager leur installation dans les lieux recevant du public. Si des initiatives sont prises localement pour installer des défibrillateurs, force est de constater qu'elles demeurent encore insuffisantes et manquent parfois de cohérence. Nous proposons d'établir une obligation d'installation d'un défibrillateur automatisé externe pour certains établissements recevant du public, ou ERP, sans préjudice de la décision individuelle d'installation d'un DAE par toute personne jugeant opportun L'installation des défibrillateurs automatisés externes au sein des établissements recevant du public, modulée selon la catégorie et la capacité d'accueil de personnes des ERP, présente un intérêt certain en termes de santé publique et a fait l'objet de recommandations par le Conseil français de réanimation cardio-pulmonaire et par l'Académie nationale de médecine, qui ont souligné l'intérêt d'installation de ces dispositifs médicaux dans les lieux de passage fréquentés par une population importante- gares, centres commerciaux, salles de spectacle où statistiquement il se produira des arrêts cardiaques, ainsi que dans les lieux où le risque de mort subite est le plus important, souvent en lien avec un effort physique- 800 sportifs sont victimes d'une mort subite chaque année, dont 10 à 15 professionnels L'objectif n'est pas de mettre un défibrillateur à chaque coin de rue, mais de favoriser un maillage pertinent et une couverture optimale du territoire en équipant les lieux publics dans lesquels les accidents sont les plus fréquents, les risques potentiels les plus élevés et le public le plus nombreux. Si l'on utilise immédiatement un défibrillateur automatisé externe chez une victime en arrêt cardiaque par fibrillation ventriculaire, les chances de survie sont les plus élevées. En effet, les taux de survie, dans les études sur les arrêts cardiaques qui utilisent la défibrillation au cours des toutes premières minutes suivant l'arrêt, sont de 85 % voire plus, contre 3 % à 5 % si l'on ne fait rien. Par ailleurs, les défibrillateurs automatisés externes sont des dispositifs médicaux dont il convient d'assurer la maintenance. À l'obligation d'installation d'un défibrillateur automatisé externe dans les établissements recevant du public est ainsi logiquement jointe une obligation de maintenance desdits appareils par les propriétaires des établissements. Ce dispositif d'urgence doit être en effet en permanence en état de marche pour permettre de sauver des vies. C'est pour cela que la maintenance est indispensable. Enfin, mesdames, messieurs les sénateurs, la constitution d'une base nationale de données relatives aux lieux d'implantation des défibrillateurs cardiaques automatisés externes sur l'ensemble du territoire est essentielle. Il faut savoir où trouver un défibrillateur en cas d'urgence. Cette base de données doit permettre à tous de géolocaliser les défibrillateurs automatisés externes à proximité du lieu d'un arrêt cardiaque afin que la personne qui appelle ces services puisse utiliser le défibrillateur conjointement aux gestes de secours, mais aussi de faciliter les opérations de maintenance de ces dispositifs médicaux. Cette base nationale que nous vous proposons d'instaurer doit être accessible aux services d'incendie et de secours et de soins d'urgence, mais aussi à d'autres opérateurs publics et privés pour faciliter l'accès de la population à ces appareils en cas d'urgence.

C'est tout l'objet de cette proposition de loi que je soutiens, car il s'agit d'une réponse forte à un problème de santé publique qui doit fédérer tous les élus. La parole

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, cher Jean-Pierre Decool, mes chers collègues,

La prise en charge des victimes est une lutte contre le temps : chaque minute représente 10 % de chances de survie en moins. Alors que le SAMU intervient en 10 à 15 minutes en moyenne, l'accès rapide et effectif à un défibrillateur que la démocratisation de son usage sont des enjeux cruciaux pour le bon fonctionnement de la chaîne de survie. Dans d'autres États dotés de programmes d'accès public à la défibrillation, les taux de survie sont bien supérieurs au taux français. Une étude américaine réalisée dans les années 2000 dans les casinos de Las Vegas, où les accidents cardiaques sont nombreux pour des raisons que chacun pourra aisément imaginer, a démontré que l'accès à des défibrillateurs utilisés par du personnel formé permet d'atteindre un taux de survie de 74 %. Les pouvoirs publics français ne sont certes pas restés immobiles face à cette question. Depuis un décret de 2007, l'utilisation des défibrillateurs automatisés externes, les DAE- comme leur nom l'indique, ils fonctionnent de manière entièrement automatisée automatisée et sont donc facilement utilisables -, est ouverte au grand public. Des dispositifs de sensibilisation, voire de formation aux aux « gestes qui sauvent » ont par ailleurs été mis en place. En particulier, un arrêté de 2009 a prévu une initiation du grand public à l'utilisation des DAE. L'enjeu demeure cependant le passage de ces évolutions réglementaires dans les pratiques citoyennes. De ce point de vue, de fortes marges de progrès existent. La sensibilisation du grand public aux gestes de premiers secours demeure tout à fait insuffisante en France, 20 % seulement de la population ayant suivi une formation. C'est évidemment trop peu. Le flou entourant les obligations des collectivités publiques et privées constitue également un obstacle majeur. En l'absence d'obligation d'installation dans les lieux publics, l'implantation des DAE repose surtout sur le volontarisme. Selon les estimations des services ministériels, notre territoire compte actuellement de 160 000 à 180 000 défibrillateurs en accès public. Par ailleurs, si l'installation des défibrillateurs, qui sont des dispositifs médicaux, est en principe assortie d'une obligation de maintenance, sa mise en oeuvre est souvent difficile du fait de la complexité de la chaîne de distribution et d'exploitation. Dans ce contexte, il est très probable qu'une large partie du parc des DAE installés sur le territoire français ne soit pas fonctionnelle, ceux-ci étant bien souvent la cible de dégradations. Il ne suffit cependant pas de sensibiliser la population à l'utilisation des DAE et d'en équiper les lieux publics ; encore faut-il qu'il soit possible, dans une situation d'urgence, d'accéder rapidement à un équipement. à l'absence d'obligation en matière d'équipement s'ajoute une absence d'obligation de recensement. Il est pourtant indispensable pour un témoin d'arrêt cardiaque de localiser le défibrillateur fonctionnel le plus proche. Cette situation est d'autant plus absurde que la plupart de nos concitoyens disposent de smartphones dont la fonction de géolocalisation pourrait sauver des vies. Face à cette carence de l'action publique, des initiatives privées ont vu le jour. En particulier, l'Association pour le recensement et la localisation des défibrillateurs, ARLoD, créée en 2008, a mis en place une base de données en ligne visant à recenser l'ensemble des DAE présents sur le territoire national, avec une implication que je salue. Cette base n'est cependant pas exhaustive : chaque jour, de nombreux défibrillateurs sont nouvellement installés, devenus hors d'usage ou déplacés, sans que ces informations fassent l'objet d'un recensement obligatoire. par ailleurs rencontré les représentants d'applications mobiles, notamment ceux de SAUV Life, proposant la géolocalisation de personnes susceptibles de porter assistance aux victimes. L'intervention de ces « bons Samaritains » formés aux gestes de premiers secours et volontaires soulève cependant un certain nombre de problèmes éthiques et juridiques, notamment en matière de responsabilité. Bien qu'il ne s'agisse pas directement de notre sujet, peut-être, dans un deuxième temps, nous préciser quelles sont les évolutions réglementaires à attendre. La présente proposition de loi, qui résulte d'une initiative et de travaux largement communs à l'Assemblée nationale et au Sénat, n'a pas l'ambition d'apporter une réponse à l'ensemble de ces enjeux. Elle vise cependant à mieux encadrer les aspects les plus matériels de ces questions, en assurant l'accessibilité effective de la défibrillation cardiaque sur l'ensemble de notre territoire. Son article 3 crée tout d'abord une obligation nouvelle d'équipement par un DAE de certains types et catégories d'établissements recevant

DAE. Je me félicite bien entendu de ces dispositions, qui permettront de clarifier l'asymétrie sur laquelle repose le régime actuel : tous nos concitoyens ont le droit d'utiliser un mais il n'existe pas d'obligation générale d'équipement des lieux publics. Cette évolution législative permettra enfin aux politiques de prévention d'avancer, si l'on peut dire, sur les deux jambes. On peut cependant s'interroger sur le périmètre des ERP qui sera retenu dans le décret. Aucune orientation générale n'est en effet prévue par le texte, mais certains lieux, vous l'avez rappelé, madame la secrétaire d'État, sont un cadre propice à la survenue d'arrêts cardiaques et devraient impérativement figurer dans cette liste : je pense aux piscines, aux enceintes sportives,

Ce coût paraît relativement limité : selon le ministère de la santé, il faudrait compter entre 1 000 euros et 1 500 euros pour l'acquisition d'un défibrillateur, et 120 euros par an pour en assurer la maintenance. Selon l'Assemblée des départements de France que j'ai contactées, les véritables inquiétudes relayées par les élus locaux portent moins sur le principe de l'obligation que sur le nombre d'équipements à installer et leur lieu d'implantation. Je considère à cet égard que le décret devra ménager des marges de souplesse afin de permettre aux élus locaux de prendre les mesures les plus appropriées en fonction de la configuration de leur territoire. L'article 3 prévoit ensuite la création d'une base de données nationale

J'en terminerai en saluant l'action et la détermination de nos deux collègues parlementaires du Nord, Jean-Pierre Decool, aujourd'hui sénateur, mais qui a rédigé le texte que nous examinons aujourd'hui en tant que député, et notre ancien collègue Alex Türk, qui se sont engagés depuis plusieurs années pour faire aboutir ce texte. Cet engagement a également pris une forme très pratique et exemplaire nos deux collègues ont en effet consacré la majeure partie de ce qui constituait alors leur réserve parlementaire à l'équipement en défibrillateurs de leur département, qui en compte aujourd'hui plus de 4 000. Je voudrais également remercier Alain Milon, le président de notre commission des affaires sociales, de m'avoir confié ce rapport sur un maillon essentiel de la chaîne de survie en cas d'arrêt cardiaque. Je vous demande donc, mes chers collègues, d'adopter sans modification cette proposition de loi. Il est de notre devoir de tout mettre en oeuvre pour encourager la citoyenneté et la solidarité de nos concitoyens dans de telles situations d'urgence. La parole

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, en Loire-Atlantique, dans une petite commune, peu importe laquelle, un adolescent de seize ans a fait un malaise cardiaque alors qu'il pratiquait sa passion sur un terrain de football. La commune, répondant à sa mission de sécurité publique, et bien que n'y étant pas obligée, s'était préalablement équipée d'un défibrillateur. Celui-ci n'a malheureusement pas fonctionné en raison d'un problème de batterie et ce jeune est mort. Rien ne dit que le défibrillateur l'aurait sauvé, mais ce dysfonctionnement ajoute évidemment à la détresse et à la tristesse des parents. Nul ne peut douter de l'engagement ni du sérieux du maire de cette commune et de son équipe, néanmoins, pour lui aussi, pour eux, c'est désormais un poids à porter, et ce même s'il n'y a pas eu de conséquences juridiques. Cet exemple a ému et interpellé les élus bien au-delà des limites de cette commune, et il y a donc de vraies attentes à l'égard de la proposition de loi que nous discutons aujourd'hui. aujourd'hui. De plus en plus d'expérimentations et d'enquêtes démontrent l'intérêt de disposer d'un défibrillateur, dans les établissements recevant du public, les ERP, notamment ceux où l'on pratique une activité sportive, car c'est là que se produisent le plus fréquemment les arrêts cardiaques. Si le décès d'un sportif de haut niveau peut faire la « une » des journaux, c'est bien dans le sport de loisir que surviennent la majorité d'entre eux. Ainsi, l'utilisation d'un défibrillateur directement disponible peut réduire le temps de délivrance du premier choc de sept à trois minutes environ, avec un taux de survie sans séquelles neurologiques très important.

Rendre obligatoires l'installation et la maintenance de défibrillateurs automatisés externes dans les ERP, lieux de passage important de populations de sexe et d'âges très divers, est un impératif. C'est le sens de cette proposition de loi, et nous nous en réjouissons. À titre d'exemple, en Loire-Atlantique sont recensés aujourd'hui dans la base de données du SDIS près de 740 défibrillateurs pour 22 230

De la même façon, créer une base de données nationale relative aux lieux d'implantation et à l'accessibilité des défibrillateurs automatisés externes sur l'ensemble du territoire va dans le bon sens. Cette loi est donc nécessaire ; elle répond à un enjeu majeur de santé publique et permettra assurément de sauver des vies humaines. Je voulais profiter de cette tribune, madame la secrétaire d'État, pour attirer votre attention sur l'enjeu de la formation aux gestes de premiers secours, mais vous avez précédé, dans votre intervention, mon interpellation.

des pratiquants de sports de loisir, celui des associations sportives, de ces millions d'enfants, de seniors, de vétérans, pour qui le risque est encore plus élevé, tous ces « sportifs du dimanche » qui s'entraînent en semaine et jouent le week-end, par passion, mais aussi pour entretenir leur santé. La grande majorité d'entre eux est encadrée par des bénévoles, souvent des parents. Or, combien d'entre eux savent reconnaître un incident nécessitant l'usage d'un DAE ? Combien d'entre eux savent le faire fonctionner ? Combien connaissent seulement le protocole à suivre en cas d'accident : qui prévenir, comment prévenir, que faire en attendant les secours, sachant par exemple que la réalisation d'un massage cardiaque est nécessaire lors de l'usage d'un défibrillateur ? Notre pays souffre d'un retard considérable dans la formation aux premiers secours alors que cette formation sauverait des vies, mais aussi, je veux noter ce point, renforcerait le sentiment de citoyenneté, la cohésion de nos sociétés, chacun se sentant ainsi un peu plus responsable de l'autre. Dans le rapport de la mission de préfiguration sur la généralisation au plus grand nombre de nos concitoyens de la formation aux gestes qui sauvent, en avril 2017, Patrick Pelloux et Éric Faure rappellent que seulement 27 % des Français sont initiés aux gestes de premiers secours. Selon la Fédération française de cardiologie, moins de 20 % des témoins d'accidents cardiaques connaissent les gestes de premiers secours. Or, quatre victimes sur cinq qui survivent à un arrêt cardiaque ont bénéficié de ces gestes simples pratiqués par le premier témoin. Nous le voyons, l'enjeu de santé publique dépasse le seul cadre de l'installation, de la maintenance et de la géolocalisation des défibrillateurs, même si ce point est important. Le Gouvernement prévoit dans son plan de prévention sur la santé de former 80 % de la population aux gestes de premiers secours.

y compris pour savoir qui va assurer la formation dans les écoles, comment mieux former les bénévoles, ceux qui ont quitté l'école depuis longtemps.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, entre 40 000 et 50 000 morts sont directement causées, chaque année, en France, par un arrêt cardiaque. C'est l'équivalent de la population d'une ville comme Albi, préfecture du Tarn, ou Charleville-Mézières, préfecture des Ardennes, qui disparaît chaque année.

en 2017 ! Or un grand nombre d'études scientifiques nous dit qu'une large part de ces 40 000 à 50 000 décès serait évitable dès lors qu'une défibrillation serait pratiquée dans les toutes premières minutes suivant l'arrêt cardiaque. Certes, depuis 2007, l'utilisation des défibrillateurs automatisés externes, les DAE, est ouverte au grand public. C'est une bonne chose, mais est-ce suffisant ? En dépit de l'implication de divers acteurs publics et privés, l'accessibilité effective des dispositifs de défibrillation destinés au grand public sur l'ensemble de notre territoire se révèle encore trop faible, insatisfaisante. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui a le mérite de proposer une réponse réaliste à cette question. L'objectif d'un meilleur taux d'équipement de DAE sur le territoire devrait ainsi être atteint. Je profite d'ailleurs de cette tribune pour faire part de la démarche positive de la SNCF, qui équipe peu à peu ses trains. Dans les TGV Lyria, un défibrillateur semi-automatique se trouve à bord des rames, installé très visiblement dans la voiture-bar. Sa présence et son utilisation ouverte à tous sont signalées au départ du train par le chef de bord. La création d'une base de données nationale relative aux lieux d'implantation et à l'accessibilité des DAE est également une disposition qui va dans le bon sens. Des applications mobiles avec service de géolocalisation sont en cours de développement et pourront permettre dans quelque temps un accès rapide à cette base de données. Parce que ces deux mesures vont dans le bon sens, je voterai cette proposition de loi. Mais ne nous leurrons pas ! Tout le monde connaît cette sentence de Confucius : « Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson ».

Bien entendu, il existe des programmes de formation aux gestes de premiers secours, programmes prévus par les textes. Mais nous savons tous ici qu'en réalité, sur le terrain, le passage de ces dispositions réglementaires dans les pratiques médicales et citoyennes continue de faire défaut. Les extincteurs méritent d'être cités en exemple, car leur technique d'utilisation a été largement diffusée. Faisons de même pour les défibrillateurs ! Aussi, madame la secrétaire d'État, je fais le voeu que le Gouvernement se mobilise sur cette question de la formation aux gestes qui sauvent et, notamment, à l'utilisation d'un DAE. Puissent des mesures réglementaires être prises pour rendre ces formations obligatoires, aussi bien dans les établissements scolaires du secondaire que dans le monde professionnel ! La parole

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, notre débat porte aujourd'hui sur une question de minutes, des minutes permettant de sauver des vies lorsque survient un arrêt cardiaque. Comme l'a rappelé M. le rapporteur, le succès de la prise en charge repose sur la limitation du délai écoulé entre le début de l'arrêt cardiaque et le recours à la défibrillation, avec des taux de survie de 70 % à 85 % dès lors qu'une défibrillation est pratiquée dans les toutes premières minutes suivant l'arrêt cardiaque. À ce jour, on compterait en France environ 150 000 DAE, défibrillateurs automatisés externes, dont le déploiement ne repose que sur la bonne volonté des exploitants et dont la localisation reste aléatoire, malgré le travail remarquable d'associations telles que AJILA et son application gratuite « Staying Alive ». Partageant ce constat, notre groupe apporte tout son soutien à la proposition de loi de notre collègue Jean-Pierre Decool, qui a précisément pour objet de réunir les conditions nécessaires à un accès généralisé aux défibrillateurs sur l'ensemble de notre territoire. Grâce à ce texte, la démocratisation de l'usage l'usage des défibrillateurs va pouvoir s'appuyer, enfin, sur le caractère obligatoire de ces équipements dans certains établissements recevant du public, ainsi que sur la déclaration de leurs lieux d'implantation. Ce nouveau cadre réglementaire sera précisé ultérieurement par décrets, aussi je voudrais insister sur quelques éléments clés à ne pas négliger dans la rédaction de ces décrets. En premier lieu, il y a la nécessité de déployer des DAE connectés. Voilà bien le seul point positif du retard pris dans notre pays : avoir à disposition des équipements connectés ou connectables. Cette technologie permet de surveiller à distance et à tout moment l'état de fonctionnement du défibrillateur, facilite la maintenance de l'appareil et réduit ainsi le risque de défibrillateurs non opérationnels. Plusieurs options de connexion existent, qu'il s'agisse de défibrillateurs directement connectés ou de modules autonomes de surveillance placés sur le support ou dans la sacoche de l'appareil. Les lieux déjà équipés de défibrillateurs non connectés pourront ainsi facilement s'adapter. Je n'y vois que des avantages. Alors, de grâce, réglementons pour le XXI siècle, pas pour le XX siècle ! En second lieu, j'attire l'attention sur les normes et l'homologation des appareils, donc des fabricants et fournisseurs. Comme nous avons pu le déplorer dans d'autres secteurs, les panneaux photovoltaïques, par exemple, l'effet d'aubaine fait naître des générations spontanées de démarcheurs peu scrupuleux. Soyons donc vigilants et anticipons. Par ailleurs, je me félicite de ce que la future base de données alimentée par les exploitants des DAE soit conçue comme accessible, ouverte et que les données soient Cela permettra aux associations pionnières qui ont développé des applications gratuites de géolocalisation de compléter et d'actualiser leurs données, pour le plus grand bénéfice de la population. Pour terminer, je souhaite insister sur un point qui n'est pas directement traité par cette proposition de loi, du moins dans la version qui nous est soumise, à savoir la formation aux gestes qui sauvent, dont la défibrillation. C'est le sens de l'arrêté du 30 juin 2017 et de l'objectif de former 80 % de la population inscrit dans le plan « priorité prévention » du Gouvernement. Il faut d'urgence accélérer la sensibilisation et la formation de toutes les composantes de la population. À défaut d'une telle mobilisation, l'objectif d'encourager les témoins d'un arrêt cardiaque à procéder à une défibrillation restera un voeu pieux. De l'avis de tous les spécialistes du secours civil, l'école doit être le lieu premier de cette sensibilisation. J'y reviendrai en présentant un amendement d'appel. Mes chers collègues, saluons de nouveau l'auteur de la proposition de loi et le rapporteur pour leur travail. Ils peuvent compter sur notre soutien.

si une défibrillation était pratiquée dans les toutes premières minutes suivant l'arrêt cardiaque. D'après les chiffres transmis, le taux de survie est alors de 85 tandis qu'il n'excède pas 3 % à 5 % en l'absence de toute prise en charge. Même si ces chiffres ont déjà été donnés, il est vraiment important de les répéter pour bien nous en imprégner. En moyenne, en France, le taux de survie après un arrêt cardiaque est de 8 %, ce qui montre donc qu'il y a une grosse marge de progression et que le recours au défibrillateur est loin d'être systématique. Plusieurs raisons peuvent expliquer une telle situation. Il y a, d'abord, le manque d'information quant à la possibilité, depuis un décret de 2007, d'utilisation des défibrillateurs automatisés externes, les DAE, par toute personne, même non médecin. le manque de sensibilisation à ce problème de santé publique et sans doute la peur, pour bon nombre d'entre nous, de mal faire, d'aggraver les choses en un moment si crucial et stressant. Au-delà de ces aspects d'éducation de la population aux gestes qui sauvent, il apparaît enfin que l'accès réel aux défibrillateurs constitue en lui-même un obstacle, un frein à une prise en charge la plus précoce possible. L'un des articles de cette proposition de loi en précisant les obligations incombant aux établissements recevant du public, les ERP, pour installer et assurer la maintenance de ces appareils. En l'absence de toute obligation légale, il semble que leur installation soit quelque peu anarchique sur l'ensemble du territoire. Cela a été dit en commission, nous serons toutes et tous attentives et attentifs à ce que le nouveau décret garantisse la généralisation effective à tous les territoires, et que certains ERP, tels que les piscines et les stades, en soient bel et bien systématiquement équipés. La maintenance est, elle aussi, essentielle, car un équipement qui ne fonctionnerait pas ou fonctionnerait mal, faute d'entretien, serait évidemment inutile. De même, la géolocalisation rapide et facile, qui plus est dans une société ultra-connectée, sera un atout déterminant. Par ailleurs, au regard de l'asphyxie budgétaire dont souffrent aujourd'hui nos communes compte tenu de la rigueur qui leur est imposée depuis des années, des dotations en baisse, je souhaiterais que le Gouvernement puisse dire, ici, que ce déploiement de défibrillateurs va être pris en charge

total sera assurément moindre au final, tant ces premiers gestes de secours éviteront des dépenses ultérieures. Madame la secrétaire d'État, pouvez-vous, au gré de ce débat, nous apporter quelques précisions sur ce point de financement ? De même, si l'utilisation de ces DAE semble relativement simple, qui, ici, peut dire qu'il serait totalement serein s'il devait s'en servir pour la première fois en cas de besoin et d'urgence ? ? Je sais que le Palais du Luxembourg est équipé de DAE, mais il ne me semble pas inutile que chacune et chacun d'entre nous, nos équipes, les agents puissent bénéficier d'une formation pour être totalement à l'aise sur leur utilisation.

En outre, et sauf erreur de ma part, je crois qu'il n'a nulle part été question de fixer une date limite quant à l'obligation d'installation, ce qui pourrait laisser le temps à chacune et chacun de s'équiper, mais sans que cela aboutisse à renvoyer cette obligation aux calendes grecques. La date du 1 janvier 2020 est-elle un objectif réaliste ? ? Pour conclure, je voudrais dire que le groupe CRCE est satisfait de la suppression de l'article 1 initial, qui prévoyait une aggravation des peines en cas de vol ou de dégradation des Ces infractions étant déjà sanctionnées par le code pénal, il ne nous paraît pas nécessaire d'être plus sévères. Là aussi, je pense qu'une plus grande sensibilisation du public, le choix de faire de ce sujet une grande cause et de développer la formation pourront éviter certains gestes d'incivilité. proposition de loi est donc d'utilité publique. Le groupe CRCE la votera, en restant bien sûr attentif, vous l'aurez compris, madame la secrétaire d'État, au contenu du décret, à son calendrier de publication, afin vraiment que la mise en oeuvre soit la plus rapide possible. La

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, minutes pour vous exposer l'avis du groupe Union Centriste sur ce texte ; huit minutes, c'est la durée moyenne d'intervention des services d'urgences préhospitaliers- rapides, mais peut-être pas assez. Tout d'abord, je tiens à saluer l'excellent travail de notre collègue Daniel Chasseing, dont le rapport particulièrement renseigné ne laisse pas de doute sur l'intérêt et l'opportunité de cette proposition de loi relative au défibrillateur cardiaque. En effet, le constat est affligeant. En France, le taux de survie à la suite d'un arrêt cardiaque inopiné est particulièrement faible 8 % en moyenne ; soit, comme cela a déjà été dit, 40 000 à 50 000 décès chaque année qui pourraient être évités.

Le retour d'expérience ne laisse donc pas de doute, la diminution de ce type de décès est strictement corrélée au déploiement des défibrillateurs. Il y a urgence à agir.

Madame la secrétaire d'État, vous le savez, mais permettez-moi de le rappeler, 70 % à 80 % des arrêts cardiaques inopinés découlent d'une fibrillation ventriculaire. Dans cette circonstance, si le massage cardiaque permet d'assurer la circulation sanguine pendant un court laps de temps, c'est le choc électrique, ou la défibrillation, qui permet le plus souvent de restaurer un rythme cardiaque normal. Je vous rappelle que chaque minute perdue en cas d'arrêt cardio-respiratoire diminue les chances de survie de près de 10 %. Les DAE, qui fonctionnent de manière autonome, délivrent des instructions orales et analysent si une défibrillation est nécessaire. Dans ces conditions, la personne portant secours n'a plus qu'à se laisser guider après avoir placé deux électrodes. Grâce à ces DAE, sauver une vie est à la portée de tous. Même avec des services d'urgences préhospitalières efficaces, dont le délai moyen d'intervention est de sept à huit minutes, la défibrillation avant l'arrivée des secours peut sauver la personne en arythmie. Il faut sept à huit minutes pour intervenir, mais nous savons que, dans certains secteurs, ce délai relève de l'utopie. Les DAE ne sont pas absents de nos territoires. Les services du ministère des solidarités et de la santé ont communiqué à notre rapporteur que 160 000 à 180 000 DAE y sont actuellement déployés. Cependant, je regrette Cependant, je regrette que le grand public ne soit pas encore suffisamment sensibilisé à l'usage de ces outils, voire aux gestes de premiers secours. Il y a un travail fort de sensibilisation à faire, notamment dans nos écoles. un peu plus de quatre minutes. Rappelons-nous que les taux de survie peuvent atteindre 85 %, dès lors qu'une défibrillation est pratiquée dans les premières minutes suivant l'arrêt cardiaque. Rappelons-nous que le délai moyen d'appel aux unités mobiles est aujourd'hui de cinq minutes. Rappelons-nous qu'effectuer des manoeuvres simples de réanimation à la portée de tous- une défibrillation cardiaque très précoce -peut faire passer à plus de 30 % le taux de survie à un mois. C'est vrai ! Rappelons-nous enfin que 70 % des arrêts cardio-respiratoires surviennent devant témoins, mais que moins de 20 % des témoins entreprennent des manoeuvres de réanimation. Pour augmenter ce taux, il faut former, bien sûr, mais aussi déployer ces instruments pour les rendre facilement accessibles, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Cette proposition de loi y parviendra, j'en suis convaincue, grâce à l'installation de DAE dans certains établissements recevant du public et à la création d'une base nationale de données relatives aux lieux de leur implantation sur l'ensemble du territoire.

de cinq minutes que je parle. Puisque, en la matière, chaque instant économisé est une vie sauvée, je n'utiliserai symboliquement pas l'intégralité du temps qui m'était réservé. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, cette proposition de bon sens appelle un vote favorable et sans réserve des sénateurs du groupe Union Centriste. La parole

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier notre collègue Jean-Pierre Decool et M. le rapporteur Daniel Chasseing du travail effectué sur ce sujet et de la qualité des auditions que ce dernier nous a proposées. Il s'agit d'un sujet essentiel et consensuel, dont le Sénat s'est emparé depuis 2006, avec Alex Türk et Sylvie Desmarescaux,

Ce texte se veut donc une réponse pragmatique à une question vitale : 50 000 de nos concitoyens meurent chaque année à la suite d'un arrêt cardiaque, alors que nombre de ces décès seraient aisément évitables. En effet, mes chers collègues, il est avéré qu'en cas d'urgence absolue l'on ne dispose que de quelques minutes pour réagir avant que le décès ne survienne.

que le comportement et les actions des premiers témoins d'une scène d'arrêt cardiaque, que le recours au massage cardiaque ainsi que la présence de dispositifs publics de défibrillation sont déterminants pour augmenter les chances de survie de nos concitoyens. Comment nous résoudre, mes chers collègues, à ce que le taux de survie observé en France à la suite d'un arrêt cardiaque n'excède pas 8 alors que, selon le Conseil français de réanimation cardio-pulmonaire, ce taux de survie peut atteindre 50 % à 70 % si des mesures simples de santé publique sont prises rapidement, notamment par la vulgarisation des défibrillateurs automatiques externes ? En les exigences en matière de formation. Les arrêts cardio-vasculaires surviennent dans 75 % des cas à domicile, dans 10 % sur la voie publique et dans 2 % au travail, et les gestes élémentaires de secours sont trop peu connus du grand public pour faire face à ces situations d'urgence. Or la meilleure des préventions réside dans la formation. Ainsi, selon les conclusions du Comité interministériel de la santé, seulement 20 % de la population française a suivi une formation aux gestes de premiers secours et seuls 50 % des élèves en classe de troisième ont bénéficié de la formation prévention et secours civiques de niveau 1 », ce qui est à l'évidence largement insuffisant devant les enjeux qui nous préoccupent aujourd'hui. L'apprentissage passe donc par la répétition des gestes qui sauvent, et ce dès le plus jeune âge. D'ailleurs, les nouvelles technologies, dont nous sommes tous très friands, peuvent se révéler un moyen peu onéreux de suppléer certaines de nos lacunes. En effet, dans notre système scolaire, par manque de temps, ces formations sont rapidement survolées dans le cadre de programmes scolaires déjà très denses. De même, les entreprises ou les collectivités locales peinent, hors obligation légale, à former des référents sécurité, capables de sensibiliser le plus grand nombre aux gestes qui sauvent. Pour ce qui concerne les défibrillateurs automatiques, ils sont très faciles à manier et un décret du 4 mai 2007 précise que toute personne sans formation particulière est considérée comme apte à utiliser ce type d'appareil. dans les situations d'urgence et de stress, une formation s'avère très utile, surtout que, depuis un arrêté de 2009, un dispositif d'initiation du grand public à l'utilisation des DAE est possible en seulement une heure. lieu, aux contraintes en matière d'accessibilité. L'installation de défibrillateurs cardiaques automatiques externes sur l'ensemble de notre territoire est une très bonne chose, à condition que les appareils soient disponibles, facilement accessibles et connus du grand public. D'où la nécessité d'être vigilants d'être vigilants sur la liste des ERP qui auront obligation de s'équiper, puis d'en assurer la maintenance. Il faudra veiller à tenir compte de la réalité de chaque territoire. Surtout, en nous fondant sur les recommandations du Conseil français de réanimation cardio-pulmonaire et de l'Académie de médecine, il est souhaitable d'installer des DAE dans des lieux de forte fréquentation, tels que gares, aéroports, hôpitaux, administrations, lieux de culte, salles de spectacles, discothèques. Pour vous rassurer, sachez qu'ici, au Sénat, il y a des défibrillateurs un peu partout.

où le risque de survenance de la mort subite est plus fréquent. Jusqu'alors, l'implantation des DAE reposait sur du volontariat. Selon les estimations des services ministériels, notre territoire compterait actuellement entre 160 000 et 180 000 défibrillateurs en accès public. L'objectif est donc de systématiser leur installation et leur entretien, afin de nous assurer qu'ils soient fonctionnels en cas d'urgence, mais également de les répertorier. Les initiatives privées, comme celle de l'Association pour le recensement et la localisation des défibrillateurs, l'ARLoD, créée en 2008, ou celle de l'application « Bon Samaritain », sont à saluer. Elles soulignent que l'usage des nouvelles technologies pour géolocaliser est une piste à creuser, afin afin de permettre la traçabilité des équipements et de faciliter la coordination avec les services de secours d'urgence et avec les institutionnels, tels que les élus locaux chargés des problématiques de santé publique et de sécurité

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je dois avouer être saisi d'une certaine émotion à l'instant où j'évoque, devant vous, la genèse et les grandes lignes de cette proposition de loi. Le hasard de la vie politique veut que ce texte, en réalité une coproduction lancée avec Alex Türk, soit un texte que j'avais déposé et défendu en 2016 lorsque j'étais député. C'est désormais avec la casquette de sénateur que je viens le soutenir aujourd'hui. Cela a été dit par plusieurs orateurs, 50 000 personnes décèdent, chaque année, des suites d'un arrêt cardiaque. Faut-il pour autant s'en tenir à ce constat ? L'homme n'a jamais accepté cette fatalité de la mort. Jadis, toutes les méthodes ont été utilisées pour réanimer ces malades aux portes de la mort : jet d'eau glacée, fer rouge sur le thorax, flagellation des pieds. En 1788, Charles Kite a été le premier à faire le pari de l'électricité pour « ressusciter les morts », selon ses propres mots. Deux siècles plus tard, le premier défibrillateur automatique a fait son apparition, en 1994. L'homme a donc inventé une machine pour surseoir à la mort. Quelle technologie fantastique ! Nul doute que, dans des décennies, cette année 1994 sera un point de repère dans l'histoire mondiale de la santé. Pourtant, mes chers collègues, notre société demeura immobile face à cette invention de génie. Comme prostrée, elle observe cette technologie, sans se l'approprier. Aujourd'hui, en France, le taux de survie est inférieur à 8 %, quand d'autres pays atteignent un taux de 74 %. Plus le secteur est équipé, plus le taux de survie augmente. C'est une réalité incontournable. Pourtant, il s'agit d'un geste citoyen très simple. Vous êtes en face d'une personne qui fait un malaise. Vous ne connaissez pas la nature de ce malaise. Peu importe, vous ne vous posez pas la question. Vous agissez. Vous disposez de quatre à six minutes pour tenter de la sauver. Il s'agit d'une urgence absolue. À défaut, les fonctions vitales sont altérées et le décès survient. Ou c'est une fibrillation et l'appareil se déclenche, ou ce n'est pas une fibrillation et l'appareil ne réagit pas. C'est la haute technologie du défibrillateur qui décide. Dès 2006, je le rappelle, Alex Türk, Sylvie Desmarescaux, alors sénateurs, et votre serviteur ont aidé à équiper de nombreuses communes du département du Nord de défibrillateurs entièrement automatiques grâce à la réserve parlementaire 4 000 appareils y ont été installés, permettant de sauver plus de cinquante vies, dont celles de certains élus locaux. L'expérience est unique en France. Le réseau s'est étoffé et renforcé, mais le nombre d'appareils est toujours trop faible sur l'ensemble du territoire. D'où cette proposition de loi déposée dans un premier temps par Alex Türk, le 1 avril 2015, mais qui n'avait pas été inscrite à l'ordre du jour du Sénat. Elle avait pour objectif de rendre obligatoire l'installation de ces appareils dans les lieux publics. Pour ma part, j'ai repris le corps du texte lorsque j'étais à l'Assemblée nationale. Ce texte a été voté le 13 octobre 2016. Dès lors, chacun comprend l'importance qui s'attache au vote de ce texte. Il constitue un pas de géant au regard du retard pris par rapport à nos voisins. C'est la raison pour laquelle je remercie le rapporteur, Daniel Chasseing, et la commission présidée par Alain Milon d'avoir validé le texte sans modification. Pour sauver des vies, il faut que ces défibrillateurs soient entretenus. C'est pourquoi nous proposons la mise en place non seulement

Je pense à la nécessité de créer une base de données épidémiologiques, pour faire avancer la recherche et comprendre l'origine de cette pathologie. La formation est également indispensable. Enfin, cela a été dit, je sais que le Sénat est équipé de défibrillateurs. Mais savez-vous, mes chers collègues, où sont les appareils ? Avons-nous été formés, nous, parlementaires, les agents

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues,

fois sur dix, ils surviennent devant témoin, mais moins de 20 % des témoins accomplissent les gestes de premiers secours. Bien conscients que ces décès pourraient massivement être évités, nos collègues députés Damien Abad et Jean-Pierre Decool, ce dernier étant aujourd'hui sénateur, nous proposent un dispositif national visant à remédier à cette situation en déployant des défibrillateurs automatisés externes aux endroits où ils apparaissent comme nécessaires. En France, le taux de survie à un arrêt cardiaque est de 5 %, tandis qu'il est quatre à cinq fois plus élevé dans les pays où les lieux publics sont équipés en DAE et où la population est formée aux gestes qui sauvent. À l'heure actuelle, le taux de réanimation sur un arrêt cardiaque est d'environ 4 %, alors qu'il est de 40 % aux États-Unis, dans les zones équipées. Malgré les innovations dans le domaine des maladies cardio-vasculaires, nous assistons à une amplification du nombre de patients. Il est important de classer ce sujet au rang des enjeux de santé publique. Aussi, je me réjouis que nous puissions en débattre aujourd'hui au Sénat. Depuis mai 2007, date à laquelle toute personne a le droit d'utiliser un DAE, on compte de nombreuses initiatives dans les territoires pour aider à l'installation de tels appareils, notamment avec le concours des départements, comme cela a été le cas dans les Hautes-Alpes, où bon nombre de communes ont pu bénéficier de cet équipement au titre de leur mission de sécurité publique. Bien qu'il n'existe pas à ce jour d'obligation réglementaire imposant aux employeurs l'installation de défibrillateurs, bon nombre d'entreprises ont également décidé d'équiper les lieux de travail et de former leurs salariés aux mesures de prévention et de secours d'urgence. Pour autant, l'implantation obligatoire de DAE dans certains locaux ne constitue pas la seule réponse pour diminuer de manière significative les 111 décès par jour.

Il convient aussi d'entretenir le matériel et de former nos concitoyens aux gestes qui sauvent. Dans le texte initial, une formation était rendue obligatoire en milieu scolaire. C'est une mesure qui allait dans le bon sens, mais qui était largement insuffisante. Si nous sommes sensibilisés, dès notre plus jeune âge, à la prévention routière par exemple, on peut regretter qu'il n'en soit pas de même pour les gestes de premiers secours. Même si les attentats ont conduit les pouvoirs publics à mener des actions, notamment en milieu scolaire, et que nos concitoyens ont mesuré à quel point ces gestes pouvaient sauver des vies humaines, ces initiatives restent insuffisantes

Nos collègues de la commission des affaires sociales sont revenus sur l'aspect réglementaire de l'article 3. Ils ont souligné, à juste titre, l'importance de la définition des ERP qui sera retenue et la clarification de la chaîne de responsabilités dans la maintenance de ces équipements. C'est un aspect important du texte, car, pour un certain nombre d'entre nous qui avons été maires, l'entretien de ce matériel entraîne un coût, notamment pour les petites communes, mais aussi des difficultés matérielles supplémentaires. En zone rurale, quel sera le périmètre des ERP retenu par le décret en Conseil d'État ? Les modalités d'application de l'obligation d'équipement doivent permettre aux élus locaux de prendre les mesures qu'ils jugent appropriées, en fonction de la spécificité de leur territoire. La possibilité qui nous est offerte de créer une base nationale de données me paraît aller dans le bon sens, mais cette cartographie doit également conduire à un dispositif pertinent et efficace à l'échelle d'un bassin de vie. S'il est indispensable que les stades, par exemple, soient équipés de défibrillateurs, une réflexion portant sur les seuils et les lieux d'implantation doit être conduite afin d'éviter des aberrations liées à une réglementation trop stricte, trop stricte, inadaptée à la configuration propre de chaque collectivité publique ou de chaque entreprise. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, ce texte pose les bonnes questions, mais n'apporte pas forcément les meilleures réponses, alors qu'il s'agit de sauver des vies humaines.

de plus de précisions sur le décret en Conseil d'État, car, pour le moment, il nous semble insuffisant pour répondre aux spécificités d'équipement des différents types de territoires. Quel

quelques défibrillateurs à l'étranger, j'ai voulu faire ma petite enquête pour savoir quel était le coût d'un défibrillateur, combien il y en avait, quelles étaient les entreprises françaises qui en fabriquaient ... Pour l'heure, aucune entreprise française n'en fabrique. L'une d'elles a annoncé tout récemment

d'un amendement d'appel. Les articles D. 312-40 à D. 312-42 du code de l'éducation prévoient, dans les établissements scolaires publics et privés sous contrat, une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours, une formation aux premiers secours ainsi qu'un enseignement des règles générales de sécurité. Si de nombreux efforts sont déployés, tant dans le premier que dans le second degré, pour déployer l'enseignement« apprendre à porter secours »,APS, la formation « prévention et secours civiques de niveau 1 et la sensibilisation aux gestes qui sauvent, il demeure nécessaire de disposer d'une évaluation quantitative et qualitative de ces dispositifs par académie, ainsi que des moyens alloués.

L'atteinte de cet objectif passe avant tout par les écoliers, comme vous l'avez très justement dit. Le plan « priorité prévention », annoncé par le Premier ministre en mars, reprend cet objectif, avec une mise en place dès la prochaine rentrée scolaire. Ce plan prévoit en même temps d'améliorer l'accès aux défibrillateurs.

Il m'a également fait savoir que la mise au point de drones défibrillateurs ouvrait de nouvelles perspectives. Alors que, en cas d'arrêt cardiaque, l'utilisation de défibrillateurs permet de sauver de nombreuses vies, ce qui a justifié la multiplication des points d'installation de ces appareils, ceux-ci sont encore difficilement accessibles, notamment lorsque les lieux où ils se trouvent sont fermés ou lorsque la victime se trouve en milieu rural, où une plus faible densité de population se cumule avec une plus faible densité d'équipement et un temps de trajet plus long pour les secours, comme l'a rappelé mon collège Bernard Le drone défibrillateur paraît être une solution séduisante, car il permettrait de surmonter les obstacles évoqués par sa rapidité de déplacement, son rayon d'action et sa disponibilité permanente.

Parmi les problématiques, il y a aussi le choix des lieux d'implantation. Dans le cas des drones défibrillateurs, ne faut-il pas plutôt raisonner en termes de maillage « géométrique » ? Mais alors, dans ce cas, qui a la responsabilité de l'installation et de l'entretien ? J'espère que toutes ces questions trouveront un jour une réponse. Quel

Pour autant, le rapport sur le plan « priorité prévention » permettra également de faire un point sur les solutions innovantes, sur un plan tant technologique qu'organisationnel, pour améliorer l'accessibilité des défibrillateurs. Je pense qu'il n'est pas légitime de cibler une solution technique plus qu'une autre dans la loi,

mais je rappelle quand même que toutes nos communes sont sous contrainte budgétaire, avec l'interdiction d'augmenter les budgets de fonctionnement de plus de 1,2 % par an.

comme nombre d'entre vous, j'ai, grâce à ma réserve parlementaire, financé beaucoup de défibrillateurs depuis une dizaine d'années. C'est grâce à ma collègue Sylvie Desmarescaux, qui m'avait soufflé l'idée,

de constater que la réserve parlementaire rendait bien service, même si beaucoup l'ont critiquée. C'était une somme de près de 1,1 million d'euros dans le département de l'Ain, pour l'ensemble des huit parlementaires, que nos collectivités se partageaient pour de l'investissement.

l'automne ? Dans la continuité du point soulevé par Philippe Dallier, je voudrais vous faire observer que nous avons une influence sur les préfets ... Si peu ! S'agissant de petites sommes demandées par les collectivités

Dans la discussion générale, la parole est à M. Jean-Pierre Decool, auteur de la proposition de loi. Monsieur Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, je dispose comme vous, très certainement, de quelques années de vie publique derrière moi, et j'observe à quel point les mentalités, les états d'esprit ont évolué. Je me souviens que, dans les années quatre-vingt, lorsque nous évoquions les problèmes des quartiers difficiles, de l'économie souterraine, des zones de non-droit, nous nous faisions traiter de « sécuritaires ». Que d'inepties essuyées !

Avec les années, les problèmes d'insécurité ont évolué et les remèdes trouvent partiellement leur source dans le progrès des nouvelles technologies. C'est ainsi que des dispositifs de caméras de vidéosurveillance, appelée pudiquement vidéoprotection - vous apprécierez la nuance sémantique ont été installés dans de nombreuses villes pour témoigner d'agressions, de vols sur la voie publique, avec les résultats que l'on connaît, pour servir les enquêtes et la recherche de la vérité. Puis la nature de l'insécurité a changé. Ce ne sont plus seulement les citoyens qui en sont victimes, mais les forces de sécurité, cette force publique qui peut être physiquement agressée, mais aussi juridiquement accusée d'insulter, de porter des coups, voire de violer lors de contrôles de police ordinaires ou lors de transports de prisonniers. Et les plaintes contre les autorités se multiplient. La police protectrice doit se protéger ! Les agents des services pénitentiaires doivent se justifier ! Les sapeurs-pompiers bénévoles ou professionnels, qui n'appartiennent pas aux forces de sécurité, doivent prévenir les éventuels dérapages, et le mot est modéré. La violente agression des pompiers en décembre 2017 à Wattrelos, dans le Nord, reste dans les mémoires. Une quinzaine d'individus agressèrent avec une violence inouïe, à l'aide de marteaux, des sapeurs-pompiers. Ces derniers étaient venus secourir ceux-là mêmes qui auraient pu être des proches des agresseurs. Nous pouvons regretter, une fois de plus, que la technologie doive se substituer à la parole, à la confiance, au bon sens des hommes et des femmes, mais c'est ainsi. La société a changé et nous devons nous adapter. Certains vont y voir une atteinte aux libertés publiques et d'autres une garantie de la sécurité. Les deux concepts ne sont pas incompatibles, et nous devons tenir compte des impératifs de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL. Quel est donc l'intérêt de ce dispositif de caméras mobiles ? Je veux être très pragmatique, très concret, en privilégiant l'efficacité sur l'idéologie, sur les partis pris. Depuis 2012, les caméras mobiles sont expérimentées par les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale dans certaines zones de sécurité prioritaire afin de garantir les conditions légales des interventions. Puis, en 2016, la loi du 22 mars relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, collectifs de voyageurs, modifiée par la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, a créé un dispositif spécifique pour l'enregistrement audiovisuel des interventions des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP. de la procédure pénale et son décret d'application du 23 décembre 2016 ont prévu un dispositif d'expérimentation pour les agents de la police municipale dans le cadre de leurs interventions. Ce dispositif avait pour objectif de mener une expérimentation de deux ans se déroulant du 3 juin 2016 au 3 juin 2018, c'est-à-dire il y a tout juste dix jours. D'après le rapport d'évaluation qui nous a été transmis, 391 communes ont participé à l'expérience, donnant lieu à l'utilisation de 2 325 caméras.

Les témoignages des intéressés expriment, sans hésitation, une sorte de cri du coeur, que je traduis en ces termes : « Ne nous retirez pas nos caméras ! » Certains affirment qu'elles devraient même être obligatoires. Pourquoi ? Quelles sont les raisons profondes d'une telle détermination ? La police ne ressent plus ce lien de confiance qui devrait être naturel. L'assermentation ? Un concept qui ne signifie plus grand-chose aux yeux de ceux qui sont considérés comme devant en bénéficier. Les personnels de sécurité n'y accordent plus de force, car ils se sentent avant tout fautifs, parfois soupçonnés. Les assermentés doivent toujours rendre des comptes et se justifier. C'est triste et ce n'est pas dans cette enceinte que nous en chercherons les origines.

S'ils ont été victimes de violences, le doute n'est plus permis. Autant la parole peut être remise en cause, autant l'image vidéo ne peut pas être contestée. Elle est authentique et parle mille fois plus qu'un témoignage écrit, qui ne frappe pas. L'image a une force dont ne dispose pas la phrase. La caméra exerce ensuite un véritable effet dissuasif : l'auteur d'une contestation exprimée avec plus ou moins de violence verbale ou gestuelle, à l'issue d'un contrôle, sait qu'il est filmé. Il aura tendance à s'incliner et à ne plus chercher la provocation. Il sait que la preuve de la vidéo ne lui permettra pas de contester les conditions de son interpellation. Enfin, et c'est le troisième intérêt du système, l'agent n'est pas obligé de déclencher la caméra. C'est en fonction du caractère plus ou moins tendu de l'intervention qu'il apprécie la nécessité ou non de déclencher le système. Un policier me rappelait que, si les caméras de télévision peuvent créer des réactions violentes, les caméras mobiles ont visiblement un réel caractère dissuasif. Alors, pour une fois que quelque chose fonctionne, tentons de l'utiliser et de l'étendre à d'autres professionnels, tels que les sapeurs-pompiers et les personnels pénitentiaires, et ce dans les règles fixées par les textes relatifs à la protection des données personnelles les images ne sont pas conservées au-delà de six mois et seul le responsable du système a accès au dispositif. Mes chers collègues, pardon pour ce catalogue de textes et d'expériences vécues. La genèse de cette proposition est simple des maires de mon département du Nord, et d'autres, souhaitaient équiper les pompiers de caméras-piétons. Ils ne se heurtaient pas vraiment à un vide juridique, mais plutôt à un flou juridique, qui les dissuadait de se lancer dans l'expérience.

: le dispositif est possible lorsque se « produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique ou celle d'un tiers », qui exclut naturellement le dispositif pour les interventions de nature médicale. Il en est de même pour les services pénitentiaires, qui pourraient disposer d'un régime spécifique d'utilisation de ces caméras.

le régime de ces expérimentations pour les mois à venir, c'est-à-dire au lendemain du 3 juin, afin de rassurer les maires et les personnels concernés. Ont-ils l'autorisation de continuer à filmer, alors que l'on sait que le temps législatif, démocratique, est parfois long, et qu'il faudra transmettre cette proposition de loi à l'Assemblée nationale dans le cadre de la navette parlementaire ? Laissons les expériences se prolonger et attendons leurs bilans pour éventuellement réajuster le cadre juridique. Pour conclure, il me semble que ce dispositif, qui n'est pas la solution miracle- nous en avons conscience -, permet à la fois de protéger le représentant de l'ordre, comme la personne qui aurait pu être abusée. abusée. L'équilibre entre liberté et sécurité est trouvé, ce qui répond aux préoccupations de la population, des forces de sécurité et des élus.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, parce qu'ils incarnent l'autorité de l'État, les agents publics sont de plus en plus victimes d'insultes, d'outrages, voire d'agressions dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Depuis plusieurs années, le nombre d'agressions de policiers et de gendarmes ne cesse d'augmenter, atteignant des niveaux préoccupants. En 2016, 687 policiers ont été blessés par arme en mission et 1 984 gendarmes ont fait l'objet d'une agression. Outre leur nombre, c'est également la violence de ces agressions qui inquiète. Tout le monde ici se souvient de l'agression effroyable d'un groupe de policiers à Viry-Châtillon en 2016. Les forces de sécurité intérieure ne sont toutefois pas les seules concernées par cette montée de violence. Alors même qu'ils assurent des missions de secours à personne, les sapeurs-pompiers sont également soumis à une agressivité croissante dans le cadre de leurs interventions. En 2016, 2 280 d'entre eux ont déclaré avoir été victimes d'une agression, soit une augmentation de 18 % par rapport à l'année précédente. Les agressions physiques commises à l'encontre des personnels pénitentiaires sont également en hausse : plus de 4 000 surveillants sont blessés chaque année dans le cadre de leurs missions. Il faut ajouter à ce chiffre les quelque 12 000 agressions verbales dont ils sont victimes. Face à ces actes intolérables, le législateur n'est pas resté inactif. Récemment, la répression des actes commis à l'encontre des agents publics a été renforcée. Depuis 2017, les peines encourues pour outrage à personne détentrice de l'autorité publique ont ainsi été augmentées et alignées sur celles encourues pour les outrages à magistrat. Des initiatives ont également été prises en matière préventive. Parmi celles-ci figure la mise en place des caméras mobiles, plus communément appelées « caméras-piétons ». Ces caméras mobiles ont été initialement mises en oeuvre à compter de 2013, et uniquement à titre expérimental, au bénéfice des agents de la police nationale. Elles ont été pérennisées pour l'ensemble des policiers et des gendarmes en 2016. Une expérimentation a été lancée, la même année, pour les agents de police municipale et les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP. L'objectif de ces caméras est double. Il s'agit, d'abord, de mieux protéger les agents contre les accusations parfois excessives dont ils font l'objet. En cas de contentieux ou de contestation des conditions dans lesquelles s'est déroulée une intervention, les enregistrements vidéo constituent des éléments de preuve objectifs, susceptibles d'être utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire. Il s'agit, ensuite, face à la dégradation des relations entre les forces de l'ordre et une partie de la population,

Dans les faits, le recours aux caméras mobiles a démontré toute son utilité. L'effet modérateur sur le terrain a effectivement été ressenti. Le simple port d'une caméra par les agents a eu un effet dissuasif et parfois permis d'apaiser des situations tendues. La proposition de loi déposée par notre collègue Jean-Pierre Decool, qu'il nous revient aujourd'hui d'examiner, vise à étendre l'usage de ces caméras mobiles à d'autres catégories d'agents de sécurité dont les conditions d'intervention se dégradent chaque jour. La commission des lois a validé, sur le principe, l'extension proposée à ces deux catégories d'agents. La protection de nos agents publics est devenue une nécessité. Les violences commises à leur égard constituent en effet une atteinte à notre République, ce que nous ne pouvons tolérer Notre commission a toutefois estimé nécessaire d'apporter plusieurs modifications à la proposition de loi, avec deux objectifs : d'une part, assurer la proportionnalité des dispositifs proposés et garantir le droit au respect de la vie privée d'autre part, adapter les dispositifs proposés aux besoins du terrain. L'extension de l'usage des caméras mobiles aux sapeurs-pompiers n'allait pas de soi. Pour la première fois, en effet, l'usage de ces caméras serait étendu à des agents qui ne remplissent pas une mission de sécurité publique.

Le nouvel article retenu restreint, tout d'abord, l'usage des caméras individuelles aux seuls cas où « se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique Il exclut, ensuite, la possibilité pour les sapeurs-pompiers de recourir aux caméras individuelles à l'occasion d'interventions à caractère médical, de manière à assurer le respect du secret médical. Compte tenu des délais de lancement d'une telle expérimentation, notamment liés à la nécessité de passer des marchés publics pour l'acquisition des équipements, la durée de l'expérimentation sera allongée de deux ans Un rapport devrait également être remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation. Enfin, la rédaction adoptée par la commission prévoit que le décret d'application de l'article sera non seulement pris en aussi après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. En ce qui concerne les surveillants pénitentiaires, la commission des lois ne s'est pas contentée de valider le dispositif proposé, elle l'a également étendu. Bien entendu, il ne s'agit pas d'étendre l'usage de ces caméras à tous les surveillants ni à toutes les missions qu'ils remplissent. Toutefois, l'usage des caméras mobiles pourrait se révéler utile dans le cadre des missions qui présentent un risque particulier d'incident ou d'évasion, soit en raison de leur nature- je pense, par exemple, aux missions des équipes régionales d'intervention et de sécurité appelées en cas de crise -soit en raison du niveau de dangerosité des détenus concernés- détenus violents ou radicalisés, notamment. Il m'a d'ailleurs été rapporté que l'administration pénitentiaire avait déjà recours à des caméras mobiles. L'extension a donc, à tout le moins, le mérite de donner un cadre à ces pratiques ! En contrepartie de cette extension du champ de l'article 2, la commission des lois a estimé préférable de rendre le dispositif expérimental pour une durée de trois ans. De plus, la commission des lois a souhaité profiter de cette proposition de loi pour pérenniser l'usage des caméras mobiles par les polices municipales. L'expérimentation, lancée en 2016, a bien pris fin le 3 juin 2018, sans que le Gouvernement ait transmis le rapport d'évaluation dans les délais impartis. Nous nous trouvons désormais dans une situation de vide juridique, qui fragilise l'usage de ces caméras par les communes. Cette situation, madame la ministre, nous la déplorons fortement, car elle place aujourd'hui les communes dans une position pour le moins complexe. Nous sommes chaque jour confrontés, sur le terrain, à des maires qui s'inquiètent de l'avenir de ce dispositif Vos services ont bien voulu me transmettre un rapport d'évaluation provisoire de cette expérimentation. Ce rapport dresse un bilan très positif de l'expérimentation conduite. Au total, 344 communes ont demandé à pouvoir se doter de ces caméras et 2 106 caméras ont été déployées. Le caractère dissuasif du port des caméras par les policiers municipaux, comme pour les forces de l'État, a été salué par la plupart des communes concernées. Face à ce bilan positif, la commission des lois a décidé de compléter la proposition de loi afin de pérenniser le dispositif. Nous espérons désormais, madame la ministre, que cette proposition de loi fera rapidement

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement se félicite que votre Haute Assemblée ait pris l'initiative d'inscrire ce débat à son ordre du jour et juge particulièrement bienvenue cette proposition de loi relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique. Je ne reviendrai pas sur la genèse des différentes dispositions législatives adoptées par le Parlement depuis 2016, qui ont progressivement étendu le cadre légal autorisant les membres des différentes forces de sécurité à utiliser une caméra mobile, qu'il s'agisse des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, des membres des forces de sécurité intérieure, puis, enfin, des agents de police municipale.

qui présente de réels atouts opérationnels et qui constitue un facteur d'apaisement des possibles tensions entre les forces de l'ordre et la population. À ce titre, dans le cadre de la police de sécurité du quotidien lancée en février dernier, avons décidé de multiplier par quatre le nombre de caméras-piétons au sein de la police et de la gendarmerie nationale afin d'atteindre le nombre de 10 000 caméras d'ici à 2019. Nous considérons qu'à terme, quand ces équipements seront largement diffusés, déclencher sa caméra, en cas d'incident ou de situation qui s'envenime, doit devenir un réflexe pour chaque policier ou gendarme affecté sur le terrain. Je n'insisterai du reste pas plus sur le fait que l'usage de cet équipement me paraît plus efficient, en termes d'apaisement des relations entre forces de l'ordre et population, que l'instauration d'une obligation de délivrance d'un récépissé en cas de contrôle d'identité. Le législateur l'avait d'ailleurs admis dans le cadre de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté en instaurant une expérimentation afin que tout contrôle d'identité fasse l'objet d'un enregistrement au moyen d'une caméra mobile. Le périmètre retenu pour cette expérimentation par le décret du 25 avril 2017 a été celui de zones de sécurité prioritaire réparties dans 21 départements. Le bilan de cette expérimentation, qui s'est achevé le 1 mars dernier, est en train d'être tiré, notamment afin d'évaluer l'impact de cette obligation sur le déroulement des interventions. Dans le droit fil des orientations retenues sous la précédente législature, le Gouvernement entend donc maintenir le recours le plus large possible, dans un cadre de sécurité publique, à ces équipements et s'emploie à les déployer. À l'origine, le but À l'origine, le but principal de la proposition de loi était- vous l'avez rappelé -de créer, à l'instar de ce qui a été prévu en 2016 pour les policiers municipaux, une expérimentation relative à l'usage des caméras mobiles pour les sapeurs-pompiers. Le Gouvernement comprend l'intention et l'origine d'une telle proposition. C'est avec la plus grande fermeté que le ministère de l'intérieur a condamné les récentes agressions, que vous avez rappelées, monsieur le rapporteur, dont ont été victimes des sapeurs-pompiers dans l'exercice de leurs missions de secours. C'est avec fermeté que de tels actes doivent être réprimés ! Et c'est avec la même fermeté que nous nous employons à faire en sorte que leurs interventions puissent s'effectuer dans des conditions optimales de sécurité, en particulier en prévoyant qu'ils soient accompagnés par les forces de l'ordre si cela apparaît nécessaire. À ce titre, la possibilité offerte aux sapeurs-pompiers de filmer leurs interventions constitue-t-elle pour eux un moyen de sécuriser ces dernières ? Le Gouvernement n'en était pas persuadé. En effet, les situations opérationnelles dans lesquelles ils sont amenés à se trouver engagés peuvent poser des questions en termes de respect de la vie privée- dans la mesure où ils sont amenés à pénétrer dans des domiciles sans mandat judiciaire -et du secret médical. Pour autant, le Gouvernement note que le travail de qualité effectué par votre commission des lois, sous la houlette de son rapporteur, aura permis d'apporter une réponse à ces questions en prévoyant que l'enregistrement ne saurait être déclenché « dans les cas où il est susceptible de porter atteinte au secret médical

ne pourra pas constituer l'alpha et l'oméga pour la sécurité des sapeurs-pompiers, et qu'il conviendra de rester particulièrement attentifs à la bonne mise en oeuvre des instructions données par ailleurs pour leur garantir un niveau de sécurité optimal. Le deuxième aspect du texte initial visait à créer un régime permanent d'utilisation des caméras mobiles, similaire à celui dont bénéficient actuellement policiers et gendarmes, par les agents de l'administration pénitentiaire chargés des missions d'extractions judiciaires ou de transfèrements administratifs. Le Gouvernement est, bien entendu, favorable à un tel dispositif. Il y souscrit d'autant plus volontiers que votre commission des lois a fort opportunément élargi le champ de cette faculté aux personnels de surveillance chargés de « missions présentant, à raison de leur nature ou du niveau de dangerosité des personnes détenues concernées, un risque particulier d'incident ou d'évasion ». Suivant la logique retenue lors de chaque extension du cadre légal d'usage des caméras mobiles, votre commission a préféré un dispositif expérimental à un dispositif pérenne, ce qui apparaît cohérent aux yeux du Gouvernement. par l'article additionnel introduit par votre commission dans le texte de la proposition de loi et qui vise à pérenniser l'expérimentation prévoyant l'usage de caméras mobiles

son démarrage à la prise d'un décret qui nécessitait la consultation de la CNIL, pour des raisons évidentes et que chacun comprend. Ce décret étant sorti à la fin du mois de décembre 2016, il en est résulté que la délivrance des autorisations et l'acquisition du matériel par les communes n'ont permis de faire démarrer réellement l'expérimentation que dans le courant de l'année 2017. difficile, au vu des textes débattus depuis le début de la nouvelle législature, de se prononcer sur l'opportunité de pérenniser ou d'abandonner une expérimentation qui venait à peine de commencer.

Deuxièmement, l'acquisition de caméras mobiles par les communes a fait l'objet d'un soutien financier de l'État, via le Fonds interministériel de prévention de la délinquance, à hauteur de 171 000 euros en 2017- 116 communes en ont bénéficié pour l'achat de 893 caméras. Troisièmement, les rapports reçus des communes ayant participé à l'expérimentation insistent sur le caractère dissuasif du port des caméras par les agents. Le constat d'une responsabilisation des personnes filmées et d'un plus grand respect envers les agents de police municipale est unanimement partagé. Les rapports précisent que le port de caméras individuelles présente un caractère rassurant pour les agents et a permis de réduire l'agressivité des particuliers, ainsi que les infractions d'outrage à agent. Des communes soulignent que, grâce au port de caméras, il a été possible d'apaiser des situations qui auraient pu dégénérer en un outrage envers les agents de police municipale. De nombreuses communes précisent, enfin, que leurs agents de police municipale n'ont pas eu l'occasion de procéder à un enregistrement. les caméras mobiles ont permis de recueillir des éléments de preuve lors de certaines interventions des agents de police municipale. À plusieurs reprises, des extractions ont été utilisées dans le cadre de procédures judiciaires et certaines ont permis d'identifier des contrevenants. Cinquièmement, plusieurs communes ont souligné l'utilité pédagogique du dispositif. Les policiers municipaux peuvent ainsi se former aux gestes et techniques d'intervention et améliorer leurs pratiques en visionnant les enregistrements réalisés lors d'interventions. Je crois donc qu'un bilan particulièrement positif peut être tiré de l'usage des caméras mobiles par les agents de police municipale, ce qui explique les nombreuses demandes de pérennisation du dispositif que nous avons reçues. Dans ces conditions, le Gouvernement soutient pleinement cette initiative, ainsi que la proposition de loi dans son ensemble. Il s'emploiera, dans le cadre d'un agenda parlementaire très chargé, à faire en sorte que ce texte, si vous décidez de l'adopter, puisse être examiné au plus vite par l'Assemblée nationale. Enfin, pour répondre à la question

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, en octobre 2015, le Comité interministériel à l'égalité et à la citoyenneté affirmait dans un rapport que l'expérimentation du port des caméras-piétons « est un succès reconnu par tous ». Il ajoutait : « Dans un contexte de violences croissantes commises à l'encontre des agents publics, le recours à l'enregistrement vidéo et sonore objective les faits en cas de recours à la coercition proportionnée. Il joue un rôle dissuasif dans la montée des tensions et aide dans de nombreux cas à prévenir le passage à l'acte violent.

Alors que le débat sur les rapports entre la police et la population, notamment dans les quartiers sensibles, a été relancé par la violente interpellation dont a fait l'objet un jeune homme à Aulnay-sous-Bois en février 2017, il semble important de rappeler que les attentes envers ce dispositif divergent, selon que l'on est un représentant des forces de l'ordre ou un citoyen. Nos concitoyens perçoivent généralement ces caméras comme un moyen d'éviter les bavures policières et les contrôles au faciès- si et seulement si -elles filment en continu. Or ce cas de figure n'est, pour l'instant, pas envisagé. Les syndicats de policiers, quant à eux, se félicitent que la vidéo ne soit déclenchée que sur l'initiative des policiers, au nom de l'autonomie sur le terrain des forces de l'ordre. C'est notamment pour répondre à ces préoccupations que plusieurs décrets ont été adoptés à la fin de décembre 2016 afin d'étendre l'expérimentation, pendant deux ans, de ces caméras individuelles par les agents de police municipale et les agents de sûreté de la SNCF et de la RATP dans le cadre de leurs interventions. Rappelons que ces décrets viennent apporter des précisions complémentaires quant aux conditions d'utilisation de ces caméras. La prévention des incidents au cours des interventions, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves et la formation des agents de police municipale sont les principaux enjeux des décrets de décembre 2016.

contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale. Le caractère dissuasif de ce dispositif a été unanimement reconnu par la direction générale de la police nationale, qui a salué « leur effet modérateur » dans les zones-test. du code de la sécurité intérieure fixe les conditions d'utilisation des caméras mobiles par les agents de sécurité. Il précise, en effet, que « dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire les gendarmes et les policiers nationaux peuvent déclencher l'équipement « en tous lieux », « lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident », après avoir prévenu les personnes filmées. Tout enregistrement permanent est donc clairement exclu. L'obligation d'information est aussi respectée avant le déclenchement de la caméra. De plus, il convient de le souligner, une fois filmées, les images ne peuvent être consultées qu'à l'issue de l'intervention et « après leur transfert sur un support informatique sécurisé ». Sauf utilité pour une quelconque procédure, elles seront effacées « automatiquement » au bout de six mois. L'utilisation de ce dispositif par les policiers municipaux a donc été réalisée à titre expérimental dans les mêmes conditions. Ainsi définies par le code des transports, les règles encadrant le dispositif pour les agents de la SNCF et de la RATP sont les mêmes.

Forts de ce bilan positif et malgré quelques critiques relatives particulièrement au droit d'accès des images filmées par les personnes concernées ou encore aux risques d'atteinte à la vie privée, nous estimons qu'il est opportun d'étendre l'expérimentation de ces caméras-piétons à d'autres agents de sécurité publique, dont font partie les agents pénitentiaires ou des sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels. Par conséquent, l'harmonisation des règles d'utilisation et le déploiement de caméras mobiles au bénéfice des agents de sécurité publique permettront notamment de s'assurer de la proportionnalité des conditions de mise en oeuvre du dispositif avec le droit au respect de la vie privée. Mes chers collègues, l'utilité et l'efficacité de ces caméras ne sont plus à démontrer dans un contexte où nos agents de sécurité publique sont confrontés à une agressivité croissante dans l'exercice de leurs missions. Nous nous devons de leur apporter un cadre juridique harmonisé afin qu'ils puissent se prémunir contre des accusations parfois excessives. Nous devons leur garantir un cadre légal qui leur permettra de se défendre correctement lors d'une procédure judiciaire. Mais n'oublions pas, afin de rassurer nos concitoyens, que les règles d'utilisation de ce dispositif doivent aussi respecter le droit à la vie privée. D'où la nécessité d'encadrer « justement » et « strictement » l'usage de ces caméras mobiles.

il reste quelques ajustements à faire pour les professions non réglementées, telles que les pompiers et les personnels pénitentiaires. J'ai donc décidé de cosigner la proposition de loi portée par mon collègue Jean-Pierre Decool afin que l'on puisse « harmoniser et aligner le régime juridique applicable à l'utilisation des caméras mobiles individuelles tout en étendant son champ d'application sous forme expérimentale ou non ». Quant au groupe du RDSE, il soutient sans réserve cette proposition de loi. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, tout récemment, alors que l'expérimentation des deux années de port de caméras-piétons par les polices municipales a pris fin, les maires des 300 communes expérimentales et des syndicats de police viennent de s'exprimer de façon unanime sur leur efficacité contre la délinquance et les incivilités. Et parmi celles-ci, on trouve deux villes de mon département, Guise et Marle. le vide juridique en ce qui concerne la pérennité du port de caméras par les polices municipales est un mauvais signe donné aux policiers municipaux et un excellent signe, si je puis dire, pour les délinquants Le rapport d'expérimentation évoqué par le ministre de l'intérieur ne nous est parvenu, par mail, qu'hier en début de soirée. Il confirme bien l'unanime satisfaction des utilisateurs. Cette proposition de loi, que j'ai cosignée, s'inscrit donc dans une suite logique de prévention des conflits, mais aussi de protection des agents en charge de notre sécurité, qu'ils soient policiers municipaux, sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, ou personnels pénitentiaires. Je rappelle que les agents chargés de la sécurité de la RATP et de la SNCF sont aussi équipés de ce dispositif, et ce depuis 2015. Il est donc temps d'en proposer un élargissement. En cet En cet instant, je souhaite évoquer la situation des personnels pénitentiaires, déjà en sous-effectif- je les rencontre régulièrement dans le cadre de la mission budgétaire « Justice » -, et visés par l'article 2. Je veux ensuite rappeler un chiffre : on recense en effet chaque année- et selon un chiffre communiqué par la direction de l'administration pénitentiaire un peu plus de 4 000 agressions déclarées de surveillants, soit plus de dix par jour -, avec une interruption temporaire de travail, pour plus de 300 d'entre elles. Parmi ces agressions, on recense 51 prises d'otages de personnels depuis 2011.

S » en raison d'une « tendance à la radicalisation », s'est évadé lors d'un transfert médical. L'homme de 21 ans a réussi à s'échapper, avec l'aide d'un complice extérieur, au moment de son arrivée au CHU de Brest, l'escorte n'étant pas- pas- ou peu -armée. Il semblerait que les escortes pour extraction médicale sont- et cela semble être su des prisonniers, en tout cas de celui-ci -sous un niveau moindre de sécurité. Il semblerait même qu'il ait

ont été récemment confrontés- et par trois fois -les personnels du pôle de rattachement des extractions judiciaires de Lille : ils ont été pris à partie par des véhicules sur l'autoroute, dans l'agglomération de Lille. Un outil de ce type aurait pu permettre une identification des auteurs. Ces personnels ne sont pas à l'abri d'une tentative d'évasion par aide extérieure. Pouvoir filmer lors d'une situation de danger immédiat constitue donc une source de preuves, vous l'avez rappelé, madame la ministre. De même, lorsqu'ils présentent des détenus devant les différents tribunaux, lesquels n'ont pas tous un niveau de sécurité adapté à leurs missions- je veux parler de l'accès des escortes, des geôles, des couloirs de circulation à l'intérieur empêchant toute personne étrangère de venir au contact -, il leur arrive souvent

que cet événement montrait « la nécessité de poursuivre et d'achever rapidement les travaux engagés pour harmoniser les règles, les procédures et les moyens mis en oeuvre pour l'ensemble des missions extérieures assurées par l'administration pénitentiaire, que ce soit des extractions judiciaires ou médicales ou des permissions de sortie sous escorte

pour objet ce que j'évoquais au début de mon intervention : il assure la continuité du port de caméras par la police municipale, dans une sorte de parallélisme des formes, et dans la suite logique du rapport d'évaluation publié hier soir.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, c'est décidément une belle journée pour notre

L'usage des caméras mobiles a été pérennisé et étendu à l'ensemble des agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale par la loi du 3 juin 2016. Son article 114 autorisait également, à titre expérimental jusqu'au 3 juin 2018, l'usage de ces caméras par les agents de la police municipale. La loi du 22 mars 2016 a, quant à elle, permis de conduire une expérimentation similaire d'une durée de trois ans, qui prendra fin le 1 janvier 2020, au bénéfice des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP. La proposition de loi de notre collègue

un renforcement de leur protection et une meilleure sécurisation de leurs interventions. Le déploiement des caméras mobiles au bénéfice des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des polices municipales a clairement démontré son utilité et son efficacité. Les caméras-piétons constituent un outil de pacification des relations entre les citoyens et les forces de l'ordre, ainsi qu'un outil de prévention des incidents. La proposition de loi soumise à notre examen fait l'objet d'un large consensus. Toutefois, la commission des lois a souhaité mieux sécuriser les dispositifs proposés ; nous partageons son initiative. Je ne reviendrai pas sur les diverses nouvelles rédactions qui ont déjà été évoquées par les précédents orateurs et, en particulier, par notre rapporteur Dany Wattebled, de manière très précise et exhaustive. Saluons seulement le le renforcement du respect de la vie privée et du secret médical, ainsi que le fait que certaines dispositions requièrent à la fois un décret en Conseil d'État et un avis motivé de la CNIL pour l'utilisation des données personnelles. Saluons

dont l'expérimentation s'est achevée le 3 juin dernier ; c'est même son premier objet. Au vu du rapport d'évaluation transmis au Parlement par le ministère de l'intérieur, le bilan de l'utilisation des caméras mobiles se montre largement positif

Les rapports sur l'utilisation des caméras transmis par ces communes au ministère de l'intérieur insistent essentiellement sur le caractère dissuasif du port de ces caméras par les agents des polices municipales. Elles permettent notamment de réduire l'agressivité de certains de nos concitoyens envers les policiers et revêtent, de fait, un caractère rassurant pour les agents de police. Face à la fin de l'expérimentation, le 3 juin dernier, les communes éprouvaient une inquiétude légitime. Nous nous réjouissons donc que ce dispositif puisse être pérennisé

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, Ce que Foucault sent, c'est que le pouvoir va devoir procéder autrement, beaucoup plus souplement, insidieusement, et en faisant une sorte d'échange : on troque une partie de notre liberté au nom d'une vie plus fluide. Il anticipe le fait qu'on passe d'un régime disciplinaire à un régime plus normatif. » C'est ce qu'explique Alain Damasio, romancier et auteur de. « On troque une On troque une partie de notre liberté au nom d'une vie plus fluide », et même si fluide que ce genre de texte ne suscite désormais plus le moindre froncement de sourcils en commission des lois. Sous couvert de pacification des relations entre l'État et ses administrés, on nous propose aujourd'hui d'étendre un dispositif jusque-là réservé aux forces de l'ordre- police nationale et gendarmerie -à d'autres agents de la fonction publique : policiers municipaux, d'abord, puis sapeurs-pompiers et agents de l'administration pénitentiaire. L'extension du dispositif à la police municipale, dont l'expérimentation vient de s'achever, présenterait un « bilan très positif », selon Gérard Collomb. Nous regrettons que le rapport d'évaluation n'ait été rendu public qu'hier en début de soirée. Au-delà

pas aborder cet après-midi. Je rappellerai que, pour notre part, nous n'étions pas favorables à cette expérimentation. Nous jugeons que sa pérennisation n'est pas souhaitable, comme nous avons eu l'occasion de le dire lors de la discussion de notre proposition de loi relative à la lutte contre les contrôles au faciès.

Se pose alors la question du but de l'opération : s'agirait-il d'avoir des éléments de preuve pour porter plainte contre son interlocuteur, sans que celui-ci puisse s'en défendre ? « Surveiller et punir », donc, puisque les images qui seront transmises aux magistrats seront celles qui seront filmées par une seule et même partie. La question du traitement des images est aussi importante : ces caméras sont souvent présentées comme un outil prétendument économique pour l'apaisement des relations entre forces de l'ordre et population, mais des moyens devront être donnés au personnel qui traitera les données filmées. Dès lors, ne vaudrait-il pas mieux consacrer ces moyens au traitement des causes profondes de la délinquance, par exemple en déployant une véritable police de proximité partout sur le territoire et en repensant notre politique carcérale ? Enfin se pose la question de la protection des données personnelles. Il est prévu qu'elles soient détruites au bout de six mois, hors le cas où elles seront utilisées dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire. Dans ces derniers cas, en revanche, nulle mention des délais. Qu'en est-il ? La vidéosurveillance « constitue le premier pilier de ce qu'on peut appeler la " société de surveillance " » : l'acuité des propos d'Alex Türk, ancien sénateur et président de la CNIL, est intacte, quoi qu'en disent les auteurs de la proposition de loi. Dans un contexte de tout-sécuritaire et de réduction des dépenses publiques, la proposition qui nous est faite ne répond pas aux inquiétudes bien réelles et légitimes des professionnels, mais comporte de multiples risques de dérives. après la police, les pompiers et les personnels de l'administration pénitentiaire, pourquoi pas, demain, les personnels hospitaliers, qui sont régulièrement pris à partie, ou encore les instituteurs ou les professeurs dans certains établissements scolaires

ne seront pas moins pris à partie avec une caméra mobile installée sur leur uniforme. Si ! Les violences à leur encontre sont bien réelles et inadmissibles, mais il ne s'agit pas simplement de s'insurger Elles s'inscrivent dans une problématique plus globale de relation distendue entre certaines populations et les représentants de l'autorité étatique, sous quelque forme qu'elle s'exerce. Multiplier le recours à la technologie dans l'espace public ne résoudra sûrement pas le problème. dans les 32 propositions formulées par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France lors de l'élection présidentielle de 2017, aucune allusion n'est faite à l'usage des caméras mobiles ; en revanche, bien d'autres préoccupations s'y font jour, comme le maintien de la proximité territoriale des secours ou encore la nécessité de compenser la disparité financière entre les territoires, source d'inégalité dans le secours. Pour les agents de l'administration notons que la disposition proposée porte sur les missions d'extractions judiciaires ou de transfèrements administratifs, sachant que les caméras de surveillance dans les établissements pénitentiaires sont déjà répandues. Encore une fois se pose la question du but d'un tel dispositif. Profite-t-il à l'amélioration de la relation entre surveillants et prisonniers ? Améliore-t-il les conditions de travail des agents pénitentiaires ?

ne sont pas dupes, d'autant que le port de caméras mobiles durant les transferts de prisonniers n'est pas leur revendication prioritaire. S'ils ne refusent pas de s'accommoder du port de ces outils,

ce texte ne fait que colmater les brèches profondes dans les relations entre l'État et ses administrés. Au lieu de traiter les causes- pourquoi un tel état de fait ? -on traite les symptômes- comment se départir des violences à un instant ? Je l'affirme à nouveau : surveillance désincarnée et suspicion généralisée ne répondront pas aux vrais enjeux de sécurité publique de notre pays. Alors, madame la ministre, notre vote sur ce texte ne sera ni un vote de rejet ni un vote d'approbation,

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, en 2016, le Parlement autorisait les agents de sécurité de la SNCF et de la RATP, mais également les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, à faire usage de caméras mobiles. Ce nouvel outil, généralement plutôt bien accueilli, alimentait toutefois certaines craintes, plusieurs de nos collègues nourrissant des doutes quant à son efficacité. Deux ans plus tard, le déploiement de ces caméras individuelles a fait ses preuves elles constituent un vecteur efficace d'apaisement des tensions et de prévention des incidents, contribuant ainsi à sécuriser les interventions des forces de l'ordre. Présentée par notre collègue Jean-Pierre Decool, dont je salue l'initiative, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui vise à étendre l'utilisation de ces caméras mobiles à deux nouvelles catégories d'agents publics. Les sapeurs-pompiers, d'abord, contre lesquels les agressions ont augmenté de 20 % en 2016 d'après l'Observatoire national de la délinquance. J'en témoigne comme élu de la Haute-Savoie, mais je sais que certains de nos collègues, dont Sylvie Goy-Chavent, élue de l'Ain, partagent aussi les préoccupations qu'expriment à la fois les pompiers sur le terrain encadrement. Les surveillants de l'administration pénitentiaire, ensuite, qui sont confrontés à une population carcérale plus nombreuse et plus violente, et à des agressions malheureusement régulières. Ces phénomènes de violence sont inacceptables, et il était absolument nécessaire de répondre à la demande de sécurisation formulée par nos agents publics. L'objectif recherché au travers de cette proposition de loi nous paraît d'autant plus légitime que les avantages liés à l'utilisation des caméras individuelles nous concernent tous : elles bénéficient évidemment aux agents dépositaires de l'autorité publique, mais aussi aux citoyens, qui pourraient sinon être victimes d'abus de droit et d'actes inappropriés. aussi aux magistrats, pour lesquels les enregistrements constituent des éléments de preuve objectifs, susceptibles de les aider dans leur travail. Cependant, une extension de l'usage des caméras mobiles aux pompiers et au personnel pénitentiaire n'était pas sans risque, en raison des atteintes potentielles au droit au respect de la vie privée. Il fallait donc concilier la protection de ce droit constitutionnellement reconnu avec la prévention des atteintes à l'ordre public.

Le périmètre du recours aux caméras a ainsi été strictement défini : toute personne filmée devra en être préalablement informée, et les caméras ne pourront pas être allumées en permanence.

La proportionnalité des dispositifs proposés est donc garantie, d'autant que plusieurs amendements adoptés en commission ont contribué à rééquilibrer la balance. Sur proposition de notre rapporteur, Dany Wattebled, que je félicite pour la qualité de son rapport, l'usage des caméras individuelles par les sapeurs-pompiers a ainsi été davantage encadré : afin de protéger le secret médical, le recours aux caméras individuelles a été exclu pour toutes les interventions à caractère Il a également été décidé que les décrets d'application de l'expérimentation seraient pris après avis motivé et publié de la CNIL, ce qui devrait nous prémunir des risques d'atteinte à la vie privée. Je m'en réjouis de nouveau. de ce texte en commission a été l'occasion de pérenniser l'utilisation des caméras mobiles par les agents de police municipale, dont l'expérimentation s'est achevée le 3 juin dernier. En l'absence de cadre légal, des centaines de policiers municipaux se sont trouvés à cette date dans l'obligation d'abandonner ce dispositif, et de très nombreux maires ont fait part de leur volonté de poursuivre une expérimentation jugée très positive.

chers collègues, le groupe de l'Union Centriste votera en faveur de cette proposition de loi, les caméras mobiles ayant fait leurs preuves dans la pacification des rapports sociaux. Rappelons-nous toutefois que ces dispositifs de vidéosurveillance ou de vidéoprotection ne pourront pas constituer l'unique réponse aux actes d'incivilité

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le vice-président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je commencerai par remercier nos collègues sénateurs du Nord, Jean-Pierre Decool et Dany Wattebled : ils nous permettent de nous pencher sur le sujet des caméras mobiles, qui intéresse beaucoup nos concitoyens, mais aussi bien des élus locaux. Cette proposition de loi et le travail du rapporteur sont guidés par la volonté de renforcer la sécurité des hommes et des femmes qui travaillent tous les jours à assurer celle de nos concitoyens. Cette volonté, le groupe socialiste et républicain la partage évidemment, d'autant que ce dispositif, rappelons-le, a été mis en place sous le quinquennat précédent. Déjà expérimenté par la police et la gendarmerie nationale à compter de 2013, il a été pérennisé pour ces corps et étendu à la police municipale, sous forme expérimentale, par la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement.

Y était introduite une expérimentation, qui s'est achevée il y a quelques semaines et qui visait à pacifier les relations entre citoyens et force de police en rendant systématique l'enregistrement lors des contrôles d'identité. À cette occasion, madame la ministre, nous avions évoqué la question du récépissé Bernard Cazeneuve et moi-même avions rejeté cette hypothèse, estimant que les caméras mobiles étaient bien plus efficaces pour les relations interpersonnelles dans des situations bien souvent difficiles. Avec cette proposition de loi, nous continuons donc sur une route entamée il y a plusieurs années, et ce avec un avantage certain, une visibilité accrue du fait des retours d'expérimentations. Je remercie M. le président de la commission des lois d'avoir respecté sa promesse en nous transmettant, même tardivement, le rapport d'évaluation de l'expérimentation des caméras mobiles par les agents de police municipale. Je peux ainsi conforter les propos des orateurs qui m'ont précédé et relever que ce dispositif est efficace. Les retours du terrain sont positifs, tout comme l'étaient les conclusions du rapport de 2016 sur l'expérimentation menée entre 2013 et 2016 par la police et la gendarmerie.

Elles pacifient d'abord les relations entre l'agent et le public. De ce fait, elles protègent des outrages verbaux les agents qui en sont équipés, et peuvent même prévenir les agressions physiques lors de leurs interventions. Elles peuvent aussi donner aux magistrats des éléments objectifs de preuve lors de procédures judiciaires. On aurait tort de classer la présente proposition de loi dans la catégorie des textes de nature communicationnelle, répondant à l'émotion légitime suscitée dans l'opinion publique par un fait divers isolé les difficultés rencontrées tant par les sapeurs-pompiers que par les surveillants de prison sont bien réelles, et elles sont croissantes. La commission des lois le souligne dans son rapport : rien qu'en 2016 le nombre de sapeurs-pompiers déclarant avoir été victimes d'une agression a bondi de 20 % par rapport à l'année précédente.

On se souvient d'ailleurs que le mouvement social des surveillants de prison survenu au début de cette année, d'une ampleur inédite depuis vingt-cinq ans, a été provoqué par une succession d'agressions à leur encontre. Aussi, l'usage de caméras individuelles est légitime. Il est efficace, mais il est aussi justifiable. Il serait hâtif de refuser tout moyen nouveau que la technologie peut mettre au service de notre sécurité, tant qu'il existe des garanties permettant de respecter l'équilibre fondamental entre sécurité et libertés individuelles. L'instauration de règles strictes pour contrôler cet équilibre est un défi majeur pour le législateur à l'époque que nous traversons. Pour y parvenir au mieux, nous devons avancer prudemment. Cette proposition de loi s'inscrit en général dans le même cadre juridique que celui des professions utilisant déjà des caméras individuelles. Les enregistrements ayant pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions, ils ne seront donc pas permanents au regard des conditions de mise en oeuvre de ces enregistrements. Les caméras devront être portées de façon apparente, ce qui garantit d'ailleurs leur effet dissuasif, et les personnes filmées devront être prévenues, dans la mesure où les circonstances le permettent, avec pour témoin un signal visuel spécifique indiquant que la caméra enregistre. Enfin, les agents équipés de caméras ne pourront accéder directement aux informations enregistrées. On peut ajouter à ces dispositions le cadre réglementaire qui sera fixé par le Conseil d'État, après avis de la CNIL, quant aux modalités de traitement des données personnelles provenant des caméras individuelles. Premièrement, seules les images issues des caméras fournies par les services sont susceptibles d'être enregistrées dans les fichiers. Deuxièmement, les images, les sons et l'identité du porteur sont stockés simultanément, et ce dernier doit justifier le cas échéant

la CNIL estime qu'au vu de la durée de leur conservation, et du fait que les traitements ne sont pas centralisés, le droit d'accès indirect aux images n'est pas effectif. Deuxièmement, la CNIL met le doigt sur la difficile interprétation de la loi quant aux cas dans lesquels l'enregistrement est possible, c'est-à-dire « lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées ». chers collègues, la notion d'incident et, plus encore, celle de risque d'incident sont éminemment subjectives, chacun l'aura bien compris. Enfin, les enregistrements peuvent être réalisés en tous lieux, sans distinction entre l'espace public et les domiciles privés. Selon la CNIL, « des des règles spécifiques devraient être prévues de manière à limiter toute atteinte à la vie privée des personnes concernées ». Nous l'avons fait dans ce texte, notamment pour les contrôles visant à des interventions médicales. Ces préconisations de la CNIL nous montrent que la réflexion sur la technique est nécessaire et qu'elle doit être encore approfondie. Il est problématique de traiter ces sujets par une proposition de loi.

Malgré ces difficultés, la commission des lois a travaillé et a apporté des améliorations importantes. La proposition de loi initiale, en se contentant d'étendre l'existant à d'autres catégories de personnel, ne donnait pas forcément de réponses aux problématiques évoquées précédemment. Des améliorations ont été apportées concernant les limites du cadre d'utilisation des caméras individuelles ; notre groupe les soutiendra. J'approuve également la modification de l'article 2

je vous incite aussi, si vous le voulez bien- vous l'avez évoqué vous-même -, à exercer une pression amicale sur votre collègue chargé des relations avec le Parlement pour que ce texte soit adopté rapidement, et de manière conforme, par l'Assemblée nationale.

au regard de l'article 45 de la Constitution. Je le regrette, parce que je crois sincèrement que cet amendement s'inscrivait dans la droite ligne de ce texte : j'entendais ainsi contribuer à sécuriser des professionnels qui risquent leur vie tous les jours pour protéger la nôtre. Cette question mérite en tout cas d'être débattue, et je ne manquerai pas de la porter plus loin à l'avenir sur le plan législatif. En conclusion, le groupe socialiste et républicain, je le répète, se félicite

Gardons cela en tête, ne rejoignons pas cet horizon, et gardons-nous de dérives orwelliennes que pourrait entraîner une logique de surveillance poussée jusqu'au bout. En 2007 déjà, la CNIL appelait à la vigilance dans son rapport annuel : « L'innovation technologique est à la fois porteuse de progrès et de dangers. Les individus sont tentés par le confort qu'elle procure, mais ils sont peu conscients des risques qu'elle comporte. » Aujourd'hui encore, c'est la vigilance face à ces risques qui doit être le mot d'ordre du législateur quand il touche à ces domaines. C'est avec cette préoccupation que le groupe socialiste et républicain votera en faveur de cette proposition de loi.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le recours aux caméras mobiles constitue un outil utile de sécurisation de l'intervention des agents publics. Moins de deux ans après sa généralisation par le législateur, le déploiement de caméras mobiles au bénéfice des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des polices municipales a démontré toute son utilité, cela a été Les difficultés croissantes rencontrées par d'autres agents publics conduisent aujourd'hui à s'interroger sur les possibilités d'extension de leur utilisation. En 2016, quelque En 2016, quelque 2 280 sapeurs-pompiers ont déclaré avoir été victimes d'une agression au cours d'une intervention, soit une augmentation de près de 20 % par rapport à l'année précédente. Cette situation conduit les sapeurs-pompiers à revendiquer, de manière légitime, un renforcement de leur protection. Quant aux surveillants pénitentiaires, ils doivent faire face à une population carcérale toujours plus nombreuse et toujours plus violente. Victimes d'agressions trop régulières, ils recherchent, de la même manière, une meilleure sécurisation de leurs interventions. Les manifestations du mois de janvier dernier en témoignent. La proposition de loi que nous examinons cet après-midi a été déposée par notre collègue Jean-Pierre Decool.

des agents de police municipale et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, à deux nouvelles catégories d'agents publics : les sapeurs-pompiers et les surveillants de l'administration pénitentiaire, qui sont confrontés, dans le cadre de leurs missions, à une agressivité croissante. En commission, les amendements proposés par le rapporteur Dany Wattebled, dont je salue la qualité des travaux, ont apporté quelques ajustements destinés à assurer la proportionnalité des dispositifs prévus. Ainsi, sur l'initiative de son rapporteur, la commission a limité le champ d'utilisation des caméras mobiles par les sapeurs-pompiers aux situations présentant un risque d'atteinte grave à l'intégrité physique des agents et a exclu la possibilité de procéder à des enregistrements en cas de risque d'atteinte au secret médical. La commission a par ailleurs prolongé d'une année la durée de l'expérimentation. Elle a prévu qu'un rapport d'évaluation soit remis au Parlement. Elle a précisé que le décret d'application devra être pris en Conseil d'État, après avis motivé et publié de la CNIL. La commission a également rendu expérimental, pour une durée de trois ans, l'article 2 de la proposition de loi relatif à l'utilisation des caméras mobiles par les surveillants de l'administration pénitentiaire, tout en étendant son champ d'application aux missions présentant un risque particulier d'incident ou d'évasion, soit en raison de la nature même des missions exercées par les surveillants, soit compte tenu du niveau de dangerosité des détenus concernés. Enfin, l'expérimentation de l'usage des caméras individuelles par les policiers municipaux a été pérennisée.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je tiens à remercier notre collègue Jean-Pierre Decool, dont la proposition de loi nous donne ici une belle occasion de parler de l'équipement de nos autorités de sécurité publique. Ce texte, dans sa version initiale, comportait deux avancées : d'une part, l'autorisation d'équiper les sapeurs-pompiers, à titre expérimental, de caméras mobiles ; d'autre part, la création d'un régime d'utilisation des caméras mobiles pour les agents de l'administration pénitentiaire. En commission, nous sommes plusieurs à avoir proposé d'élargir le champ d'application de ce texte. Je rappelle que l'expérimentation de deux années permettant aux polices municipales d'utiliser leurs caméras mobiles a pris fin le 3 juin dernier, dans une indifférence générale regrettable.

sur la sécurité routière, le 5 juin dernier, j'ai longuement développé les raisons pour lesquelles la pérennisation du dispositif pour nos policiers municipaux ne comportait que des avantages. Je me réjouis du vote de ces amendements, car ils répondent à une attente très forte de nos maires et de nos élus délégués. C'est pour des raisons similaires que je tiens à expliquer aujourd'hui pourquoi nous devons expérimenter l'utilisation des caméras individuelles par nos pompiers.

parce qu'ils représentent l'autorité, parce qu'ils travaillent de concert avec la police et la gendarmerie. La conséquence en est, mes chers collègues, que le nombre des agressions dont sont victimes nos pompiers explose, année après année.

peuvent être aussi urbaines. Nous savons que certains quartiers sont gangrenés par les trafics, les incivilités et la violence. Ces comportements sont le fait de petits voyous Ce sont ces voyous qui caillassent nos pompiers. Ce sont ces voyous qui crachent sur nos pompiers. Ce sont ces voyous qui s'en prennent physiquement à nos gendarmes et à nos forces de l'ordre. Alors, oui, madame la ministre, nous devons équiper nos pompiers de caméras-piétons, dans la mesure où elles remplissent deux fonctions essentielles. La première fonction est préventive. Je rappelle qu'elles sont portées de façon apparente et qu'un signal lumineux indique que la caméra enregistre, déclenchée par l'agent qui la porte selon les circonstances. La seconde fonction est de favoriser la sanction. En effet, visionner la scène est un moyen de preuve efficace dans les prétoires. Cela implique toutefois, madame la ministre, que le Gouvernement revienne sur les lois Taubira qui ont affaibli l'institution judiciaire. Cela implique aussi qu'un voyou condamné à une peine de prison ferme aille en prison ! Jusqu'à présent, vous avez beaucoup usé de paroles, mais les actes ne sont pas encore au rendez-vous ! Si vous proposez de doter la justice de moyens juridiques et matériels suffisants, croyez-moi, tous les sénateurs Les Républicains seront derrière vous- et ils ne seront d'ailleurs pas les seuls. Pour conclure, je renouvelle mon soutien aux métiers du service public de la protection, de la sécurité et de la défense. Ils incarnent l'esprit de la République et les valeurs de la France portées au plus haut. Nous avons ici une occasion très concrète d'aider ces héros du quotidien qui, pour beaucoup, sont bénévoles. C'est l'honneur du Sénat de donner à ceux qui défendent nos valeurs les moyens de réaliser leur action.

En effet, l'expérimentation de caméras-piétons pour les policiers municipaux s'est achevée le 3 juin dernier. Faute de base légale, les policiers municipaux ne peuvent donc plus utiliser ces outils depuis le 4 juin. Or, après deux ans d'expérimentation, la réussite la réussite de ce dispositif fait l'unanimité. Les caméras permettent d'apaiser les tensions, de sécuriser les missions des policiers en limitant les risques de comportement agressif, d'apporter la preuve du bien-fondé d'une intervention. Ce dispositif vise aussi bien à protéger les agents qu'à constituer des éléments objectifs de preuve en cas de litige. Il participe à la protection des citoyens et du service public. J'ai été corapporteur avec mon collègue François Bonhomme d'un rapport d'information sur la sécurité dans les transports terrestres face à la menace terroriste, qui a fait évoluer la loi Savary.

Depuis sa mise en place au mois de février 2018, ces agents peuvent enregistrer les interventions qu'ils réalisent dans l'exercice de leurs missions, au moyen de caméras individuelles.

Dans sa propension illimitée à tout compliquer et réglementer, l'État nous contraint à légiférer aujourd'hui. L'exemple des caméras-piétons en est une parfaite illustration. En France, tout le monde a le droit de filmer. Seule la diffusion publique est réglementée selon le droit à l'image. Or nous, les maires, n'avions pas attendu ni même demandé d'autorisation à l'État pour équiper nos policiers municipaux.

pour faire taire les mises en cause injustifiées. L'expérimentation a été immédiatement concluante. Les caméras protègent bien les policiers municipaux contre les mises en cause injustifiées.

Jamais un juge n'a refusé ces images au motif de l'absence de base légale ; d'ailleurs, les juges acceptent les images prises par la partie adverse. Mais voilà, pour l'État, gendarmes et policiers seraient des sous-citoyens, seuls à ne pas pouvoir filmer sans autorisation expresse et caméra homologuée. En 2016, le Gouvernement a tenu à donner un cadre légal à cet usage qui n'avait rien d'illégal. La loi du 3 juin 2016 autorisait expressément l'usage

non de prolonger l'expérimentation que l'on savait concluante bien avant que l'État ne la lance, puisque nous l'avions mise en oeuvre depuis longtemps. La caméra est aussi le meilleur régulateur de la relation police-population. C'est d'ailleurs confirmé par le rapport d'évaluation du ministère de l'intérieur en date du 7 juin

La caméra est la solution de remplacement au récépissé de contrôle d'identité, qui ne ferait qu'ajouter de la paperasse à la paperasse. Oui, il faut aussi équiper les sapeurs-pompiers, de plus en plus victimes d'agressions de la part de voyous. Le Sénat a d'ailleurs relevé

de l'administration pénitentiaire. Les premières zones de non-droit en France, ce sont non pas les quartiers, mais les prisons : surpopulation carcérale, moyens insuffisants et autorité disqualifiée par l'impunité, dans la mesure où des gardiens peuvent être insultés et provoqués à longueur de journée. La vidéo existe en prison, dans les couloirs, mais sans le son. Il faut l'image et le son pour appuyer les procédures disciplinaires et judiciaires et commencer à rétablir le droit dans ces établissements. C'est pourquoi la commission des lois a enrichi ce texte. Nous savons que les communes, pour les polices municipales, et les départements, pour les SDIS, sauront équiper leurs personnels selon leurs besoins. Nous aimerions avoir la même

plutôt que ralentir celui des collectivités. En attendant, l'adoption de ce texte est indispensable. C'est pourquoi le groupe Les Républicains le votera avec enthousiasme.

La loi de 2013 a rendu incompatible le mandat de conseiller communautaire avec un emploi salarié au sein de l'une des communes membres. Or le mandat de conseiller municipal au sein de l'une des communes membres n'est pas, lui, incompatible avec un emploi salarié au sein de l'intercommunalité. Il s'agit là d'une inégalité flagrante, qui ne repose sur aucune considération d'intérêt général.

avis défavorable. C'est par parallélisme que le législateur a introduit une règle d'incompatibilité selon laquelle l'élu communautaire, étant en même temps élu municipal, ne peut être salarié de l'une des communes membres.

si vous en acceptez le principe, de travailler à l'uniformisation des règles d'incompatibilité en les appréhendant de manière globale dans le cadre du chantier sur le statut de l'élu local que le Président de la République a indiqué vouloir ouvrir lors du Congrès des maires de France. Votre réflexion pourra ainsi utilement s'inscrire dans le cadre des travaux

Il faut essayer d'accorder aux élus un minimum de sécurité juridique. Actuellement, le fait d'être dépositaire d'une autorité est systématiquement une circonstance aggravante, jamais atténuante,

est considérée comme un délit, le délit de favoritisme. L'objet de cet amendement est d'introduire la notion d'intentionnalité-

qui ne saurait être analysée, le cas échéant, que dans le cadre d'une réflexion plus générale sur le régime de responsabilité des élus. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Arnaud de Belenet. Cet amendement vise à supprimer l'article 21 , qui a été introduit en commission. Cet article permet à un EPCI de participer à un groupement de commandes- cela ne pose pas de problème -si ses statuts le prévoient, quelle que soit par ailleurs la compétence de l'EPCI.

dans des conditions de majorité qualifiée ne permettent pas davantage de déroger à l'attribution des compétences. Contrairement aux compétences dont la liste doit figurer dans les statuts, la précision consistant à indiquer que l'EPCI pourra participer à un groupement de commandes ne mentionnerait pas

qui s'oppose à ce qu'un EPCI agisse hors des compétences qui lui sont attribuées et qu'il passe des marchés pour l'exercice des compétences qui relèveraient des communes membres. Les statuts de l'EPCI qui sont soumis aux conseils municipaux dans des conditions de majorité qualifiée ne permettent pas davantage de déroger à l'attribution des compétences. Contrairement aux compétences dont la liste doit figurer dans les statuts, la précision consistant à indiquer que l'EPCI pourra participer à un groupement de commandes ne mentionnerait pas forcément les champs sur lesquels porteront les groupements de commandes. Afin de préserver la lisibilité de l'action publique locale, il est donc nécessaire que les EPCI ne jouent pas le rôle d'acheteur au titre de compétences relevant seulement des communes.

de Mme la ministre. Je rappelle que la loi précise déjà qu'il est possible de mettre en place des services communs entre communes et communautés de communes hors de tout transfert de compétences. Je ne vois donc pas pourquoi il ne serait pas possible,

doit venir des territoires. Je rappelle que les conférences des maires servent justement à déterminer en quoi les communautés de communes peuvent leur venir en aide. C'est typiquement grâce à ce type d'article qu'on libère les énergies et que l'on permet aux communes de faire des économies substantielles.

à l'occasion de l'application de la loi sur le non-cumul des mandats. S'il y a un dispositif qui trouve toute sa pertinence et je dirais même qu'il est urgent

à Mme Catherine Di Folco. La loi MAPTAM a conduit à la création d'EPCI de taille très importante, incluant un grand nombre de communes et prenant la forme de communauté d'agglomération, de communauté urbaine ou de métropole.

à détourner ces EPCI de leur mission et génère un sentiment profond de dépossession des maires vis-à-vis de leurs administrés. En conséquence, cet amendement vise à restreindre la compétence de la communauté urbaine et de la métropole à la voirie principale, déterminée d'intérêt communautaire ou métropolitain par l'organe délibérant. Le sous-amendement

Fort utilement, il vise à restreindre la compétence obligatoire à la voirie d'intérêt communautaire dans les communautés urbaines et les métropoles. En effet, avec ces transferts, les mairies sont aujourd'hui dépossédées de cette mission essentielle de proximité qui nécessite pourtant une grande réactivité. Qu'observons-nous, madame la ministre ?

En référence à une discussion que nous avons eue hier, j'indique que nous avons dès le départ installé des pôles de proximité. La compétence « voirie » est bien évidemment exercée à l'échelle de la métropole, mais les équipes de proximité sont dans ces pôles ; ainsi, lorsqu'il y a un nid-de-poule, le maire de la commune appelle le directeur du pôle de proximité

la première année d'application des dispositions de l'article 1522, le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne peut excéder le produit total de cette taxe tel qu'issu des rôles généraux au titre de l'année précédente L'esprit de ce texte, qui ne prend pas en compte la situation des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés, est que l'instauration d'une part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, ou TEOM, ne doit pas être un moyen d'accroître le produit global de cette taxe. La conséquence collatérale de ce texte est que, en cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, l'instauration d'une TEOM avec part incitative sur l'ensemble du territoire devient impossible lorsque l'un des EPCI fusionnés avait supprimé cette taxe pour la remplacer par une redevance d'enlèvement des ordures ménagères, Ce cas n'a pas été envisagé par le législateur, puisque, hors cas de fusion d'EPCI, un EPCI n'a aucune raison de passer de la redevance à la taxe avec part incitative. Le cas de la fusion d'EPCI n'ayant pas été imaginé par le législateur, il convient de permettre le passage à la taxe avec part incitative sur l'ensemble du territoire d'un EPCI dont une partie du territoire était passée au système de la redevance préalablement à la fusion. Le présent amendement vise à insérer un alinéa supplémentaire dans l'article 1636 B 1636 B du code général des impôts afin de prévoir explicitement ce cas. Conformément à l'esprit du texte, le produit total de la taxe avec part incitative ne devra pas excéder la somme des produits des taxes et redevances des différents EPCI fusionnés.

est effectivement très technique. Cet amendement vise à permettre aux EPCI issus de fusions d'instaurer sur l'ensemble de leur territoire la part incitative de la TEOM dès la première année, y compris si un ou plusieurs EPCI préexistants avaient institué la REOM. Une telle

La présente proposition de loi n'est pas le véhicule législatif adéquat pour modifier les modalités de fixation d'une imposition locale. J'appelle votre attention sur le fait que, dans le cadre de la refonte de la fiscalité locale et dans le cadre de la feuille de route sur l'économie circulaire, le Gouvernement examine différentes évolutions juridiques relatives à la TEOM. outre, l'instauration d'une part incitative de la TEOM sur le territoire d'un EPCI nouvellement constitué pose un certain nombre de difficultés techniques.

elle ne saurait servir de base pour fixer le montant maximal de la part incitative de la TEOM dans le cadre que vous proposez. Pour toutes ces raisons, même si je comprends bien le fond du problème, je crois qu'il serait judicieux de retirer votre amendement afin de poursuivre le travail sur ce sujet dans les deux cadres que j'ai évoqués.

à M. le rapporteur. Il s'agit, là aussi, d'un sujet maintes fois évoqué par une immense majorité de maires. Cet amendement a pour objet de renforcer la sanction en cas de retard pris par l'État dans la notification aux collectivités territoriales et à leurs groupements du montant de leur attribution individuelle annuelle au titre de la dotation globale de fonctionnement. Tout retard serait présumé porter préjudice à la collectivité territoriale ou au groupement concerné jusqu'à preuve contraire.

la compétence en matière d'urbanisme pour la délivrance des certificats d'urbanisme, des permis de construireet d'autres documents a été transférée de l'État aux maires. C'était un acquis de la décentralisation. Le ministre de l'intérieur de l'époque, Gaston Defferre, a aussitôt constaté que les 36 000 communes de France n'avaient généralement pas les moyens d'exercer cette compétence. Il a donc sagement mis les services de l'État à la disposition des maires.

tiré le tapis sous les pieds des maires, leur retirant la possibilité que les services de l'État, dont les effectifs diminuaient, puissent continuer à instruire les demandes de permis de construire. En vérité, cela a induit pour nos communes une charge nouvelle et brutale au moment même où les dotations étaient drastiquement réduites et alors que des charges nouvelles étaient insidieusement transférées par l'État aux collectivités territoriales. Il me semble que, lorsque l'on représente l'État, on ne peut pas à la fois augmenter les charges des collectivités et refuser que celles-ci trouvent les financements nécessaires pour assumer ces charges. Il s'agit d'une contribution modeste qui est demandée aux usagers

la ministre, je suis convaincu, vous connaissant, et me souvenant de la présidente de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales que vous avez été, mais voyant aussi à l'oeuvre la ministre chargée des libertés locales que vous êtes aujourd'hui, que, à la lumière du débat et des échanges que nous avons, vous ne pouvez que faire évoluer votre avis pour que celui-ci vaille engagement du Gouvernement à régler ce problème en faveur de nos communes. La parole est

L'année dernière, les subventions ont été distribuées au mois de février sans que personne ait été informé de quoi que ce soit. Cette année, nous n'avons même pas été invités

coupés du terrain. Est-ce la volonté de ce gouvernement d'avoir des élus hors sol ? Telle est la question qui se pose aujourd'hui

Quatrièmement, nous avons donné des instructions très précises à tous les préfets pour que les parlementaires soient informés de l'ensemble des dossiers présentés.

Selon le code général des collectivités territoriales, « constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune Héritage de l'histoire, la section de commune a essentiellement une fonction patrimoniale. Elle possède la personnalité juridique. La gestion des biens et des droits attachés à la section est assurée en principe par le conseil municipal et par le maire. Cette gestion peut être assurée aussi par une commission syndicale élue par les habitants. Force est de constater que la complexité du régime juridique, dans la ligne droite d'un dispositif issu du droit médiéval, pose aujourd'hui de sérieuses difficultés à de nombreuses communes rurales. L'aspect de démocratie locale tend à s'estomper derrière des considérations de défense d'intérêts particuliers. L'obsolescence du cadre juridique constitue également une source de contentieux. Aussi la lourdeur de ces sections de commune suscite-t-elle des interrogations quant à leur maintien. Dans ce contexte, il est proposé de limiter les cas de création d'une commission syndicale, d'instaurer une taxe communale pour la gestion des sections de commune et de permettre au conseil municipal de prononcer la dissolution d'une section de commune selon des cas définis. Il faut bien reconnaître que, à l'heure de la construction européenne, ce principe semble tout à fait obsolète.

la prise en compte par les statuts des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la participation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à ces associations.

dont je rappelle qu'il est, en zone de montagne, de 5 000 habitants. Je pense que cette mesure créera des difficultés sur le terrain. Il en va de même pour l'exercice territorialisé des compétences : alors que, aujourd'hui, on peut organiser la proximité dans la gestion d'une intercommunalité, la mesure inscrite dans la

Ce grand saut dans le vide a suscité, partout où je passe, une organisation administrative et un fonctionnement territorial qui s'apparentent à une construction byzantine. Depuis lors, évidemment, il n'est plus question de grand soir, fût-il révolutionnaire, ni de grand meccano institutionnel, tant notre équilibre institutionnel est sorti fragilisé, et même contusionné, de cette réforme territoriale. Madame la ministre, j'ai été interloqué, hier, lorsque vous nous avez accusés de remettre en cause le principe de stabilité institutionnelle réclamé par les élus et de contrevenir

Le scrutin est ouvert.